La séance est ouverte. De compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Nous n'avons pas reçu d'observation. Il y en a-t-il en séance. Je ne vois point. Le procès verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. Madame, la Première ministre, mesdames et messieurs les Ministres, mes chers collègues. Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Notre séance et retransmise en Direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Chacun sera attentif. Au respect, à la fois du temps de parole et des uns et des autres. Je donne immédiatement la parole au président Patrick Kanner pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci président, madame, la Première ministre en préambule à ma question je rappelle un principe intangible. La violence ne peut en aucun cas être une réponse à un mécontentement social ou politique. Aussi au nom de mon groupe, je condamne l'agression dont a été victime, Jean-Baptiste Trogneux et lui apporte notre total soutien. Je manifeste le même soutien Yannick Morez, maire de Saint-Brevin-les-Pins qui a subi intimidations harcèlement et agressions. Autant d'actes inqualifiables envers un élu de la République qui ne faisait qu'exercer son mandat il mérite également mes chers collègues, le respect, le soutien indéfectible du Sénat. Oui, mes chers collègues. Un vent mauvais souffle sur notre pays. Un maire de France a dû céder devant la menace, la violence, la haine, l'a emporté sur la bienveillance la force l'a emporté sur le droit. La multiplication des pressions des agressions envers les élus et quantifiable et documenté. Les élus locaux et plus particulièrement les maires sont les fondations de la République quand une de ces fondations s'écroule comme avec la démission Edith Morel. C'est tout l'édifice qui est fragilisé. L'audition émouvante de ce dernier ce matin par la commission du le 7 du des lois du Sénat s'est transformé en réquisitoire contre les services de l'État tentes ont été révélé de graves défaillances. C'est un échec. Madame, la Première ministre pour ne pas dire un désastre dont il faut tirer toutes les conséquences des aujourd'hui. Saint-Brévin. C'est aussi le signe d'une résurgence des violences de l'extrême droite depuis plusieurs semaines. Ces actes de terrorisme intellectuel et physique se sont multipliées pour empêcher les maires qui le veulent de prendre part à l'accueil des demandeurs d'asile. Madame, la Première ministre on ne peut mettre sur un pied d'égalité l'extrême droite et d'autres formes de contestation l'extrême droite, que ce soit au sein de nos institutions ou dans le cadre d'actions clandestines et l'ennemi mortel de notre démocratie, l'État ne peut rester l'arme au pied, face à ces menaces. Allez-vous engager ce combat pour défendre les élus de la République. On vous réponde. La parole est à madame la Première ministre vous avez la parole. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, Patrick Kanner. Depuis des semaines Yannick Morez. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins. A été victime d'une campagne insupportable de harcèlement en lien avec un projet d'implantation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans sa commune Son domicile a été incendié. Alors oui ces actes sont inadmissibles. Derrière chaque élu agressé, c'est la République qui est visé. Avec chacun de vous et en évitant toute polémique. Monsieur le Président Kader. Je partage le choc et l'indignation face à cette situation comme face à chaque acte de violence contre les élus. En présentant sa démission Yannick Morez a pris une décision difficile en son âme et conscience. Nous ne pouvons que regretter qu'il ait été conduit à faire ce choix. Et naturellement, nous le respectons. Je le recevrai tout à l'heure avec l'Association des maires de Loire-Atlantique et l'Association des maires de France. Mon objectif est de l'écouter et de lui exprimer le soutien de mon gouvernement. Les maires sont en première ligne sur le terrain. Ils sont les premiers témoins de la montée de la défiance dans notre société. Nous devons les protéger. Nous devons protéger tous les élus pour y parvenir, le gouvernement s'engage. Le ministre de l'Intérieur, les préfets et les forces, les forces de l'ordre sont mobilisés. Le droit pénal a été renforcé pour permettre aux associations d'élus et aux collectivités de se constituer partie civile. À plusieurs reprises le ministre de la Justice a demandé au procureur des réponses fermes rapide visible contre les atteintes aux élus. Et nous sommes prêts à travailler avec vous comme avec l'Assemblée nationale pour renforcer les sanctions pénales contre les violences envers les et du et nous voulons aller plus loin. Depuis des mois, nous préparons des mesures nouvelles que la ministre chargée des collectivités territoriales. Dominique Faure présentera tout à l'heure, il s'agit de renforcer le lien entre les maires et la justice. De mieux prévenir les violences et d'accompagner encore davantage les élus. C'est un sujet auquel je tiens particulièrement et que j'avais eu l'occasion d'un d'évoquer avec l'ensemble des associations d'élus le 12 avril dernier. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Il n'y a pas de démocratie sans respect des élus. Pas de démocratie sans sécurité. Pour les élus, avec vous tous avec le gouvernement, nous continuerons à agir. Je vous remercie. Quelques secondes. Il demande. Qui de l'action et qu'ils puissent agir eux-mêmes et quand Madame Dominique Faure évoque la création d'un centre d'analyse pour savoir ce qui se passe dans le pays. Permettez-moi de vous dire que nous le savons depuis bien longtemps que tout est quantifié et quantifiable et que nous demandons simplement que la réflexion qui est menée, notamment au Sénat puisse être appliqué pour protéger les élus de la République. La parole est à notre collègue Véronique Guillotin pour le groupe du Rassemblement démocratique et Social Europe. Oui alors il avait la parole. Merci monsieur le président, madame, madame, monsieur, madame, madame la Ministre, avec mes collègues Jean-François Husson et Véronique Del Fabbro je vous interpelle sur les faits qui se sont déroulées samedi à Villerupt en plein centre-, ville à 2 pas d'un parc pour enfants, une fusillade a eu lieu sur fond de trafic de drogue. Le bilan humain et la violence des faits ont profondément choqué et bouleversé les habitants 5 blessés, trois dans un état grave. Tous étaient âgés entre 17 et 30 ans. Mes pensées vont bien sûr aux victimes, à leurs familles à toutes les villes russes siens et toutes les villes russes tiennent à qui nous devons apporter des réponses. Tout le monde est choqué. Mais personne ne semblait surpris. Or ce point de deal avait pignon sur rue depuis des mois, les tarifs des stupéfiants sont encore inscrits sur les murs à côté d'une fresque d'enfants. Ce drame mais effectivement lumière le débat récurrent du sous-effectif chronique de la circonscription de police. Selon lui, ville rue il manque à ce jour 15 policiers au moins vendredi le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture de 11 postes. Si cette nouvelle part d'une bonne intention, il y a peu de chances que ces postes soient pourvus par défaut d'attractivité du territoire. Madame la Ministre ce qui s'est passé est grave suite aux échanges que nous avons eu ces derniers jours avec le cabinet je salue l'arrivée d'un escadron de gendarmes mobiles dès cet après-midi à Villerupt. Pour autant, à moyen terme et afin de remonter les effectifs comptez-vous nous affecter des policiers en sortie d'école. Enfin un dernier regret la Villerupt que je suis n'a jusqu'ici pas réussi à convaincre les élus locaux de la nécessité de se saisir de tous les outils contrat local de santé police municipale vidéoprotection. Je crois que que c'est tous ensemble, pas en opposant les uns aux autres. C'est tous ensemble en laissant tomber les idéologies que nous ferons reculer la délinquance. La mise en place d'une réunion de concertation locale en urgence s'impose. Il y va de la sécurité et de la tranquillité des habitants. Je compte sur le ministre, car il est encore temps d'enrayer cette spirale infernale. J'en suis convaincu.

Pour plusieurs coups de feu tirés dans le centre-ville de Villerupt Villerupt en Meurthe et Moselle. Sur place, les policiers découvrent 5 blessés par balles, dont trois sont en urgence absolue. D'après les premiers éléments cette tentative d'homicide serait en lien avec. Le trafic de stupéfiants dans le cadre d'une recrudescence de la violence entre bandes rivales pour le contrôle de ce trafic, quelques heures après les faits, l'auteur présumé de la fille de la fusillade. Il a été interpellé par la police judiciaire de Metz assisté par la BRI. Je tiens ici à remercier tous les policiers pour leur mobilisation et leur action rapide et efficace, sur instruction de Gérald Darmanin, un escadron de gendarmerie mobile, soit 70 gendarmes. Vous l'avez dit a été envoyé sur place dès hier. au moins jusqu'à la fin de la semaine pour la circonscription de police dont dépend Villerupt. Le ministre de l'Intérieur annonce l'ouverture, vous l'avez dit aussi de 11 postes. Par ailleurs, 44 nouveaux postes seront ouverts sur l'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle. Nous constatons que le trafic de drogue touche aujourd'hui. Les villes de taille moyenne comme la vôtre. C'est pourquoi nous devons lutter contre ce trafic à tous les niveaux. Je pense à l'excellent travail réalisé par les policiers des Yvelines qui ont effectué une saisie record de 2 tonnes 5 de cannabis pour une valeur marchande de 20 millions d'euros. Il y a seulement quelques jours. Je sais que tous les élus concernés sont particulièrement mobilisés sur le sujet est particulièrement vous les sénateurs Husson Jacquin Del Fabbro et vous-. Même madame la sénatrice. Pour cette raison et vous l'avez indiqué le préfet va réunir l'ensemble des élus concernés dans les plus brefs délais. Cette réunion est d'ores et déjà programmée. Je vous remercie. Quelques secondes madame Guillotin. Oui, quelques secondes pour dire qu'effectivement quand on voit un tel drame, et qu'on entend dans la rue dire que que ça n'étonne en fait quasiment personne. Je crois qu'il y a des vraies leçons à prendre. L'État doit assumer ses responsabilités, l'État ne doit pas défaillir mais c'est main dans la main, État, élus locaux que nous devons travailler et faire reculer cette délinquance. Merci la parole est à notre collègue Ronan Dantec. Pour le groupe écologiste solidarité et territoires. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre Yannick Morez a démissionné et il ne reviendra pas sur sa décision. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins est ainsi devenue depuis quelques jours le symbole des difficultés des élus locaux à exercer leur mandat. Non plus seulement à portée d'engueulade, mais bien de calomnie d'agression aussi et dans ce cas d'un attentat criminel qui aurait pu le tuer sa femme et lui. une mauvaise n'a pas démissionné par peur ou par lassitude. Il a démissionné parce que l'État ne l'a pas protégée, il y a ni mauvaises depuis l'incendie de sa maison. Le 22 mars était devenu le symbole du courage de l'élu républicain, celui qui assume sans faiblir, la tâche que lui a confié l'État en l'occurrence le déménagement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile un Cada déjà installé sans problème dans la commune depuis 2016. Il est en tribune et c'est d'abord à ce titre que nous lui rendons hommage il tenait bon face à la haine de l'extrême droite et des sbires Éric Zemmour.

Monsieur le Ministre qu'il n'y ait pas de faux débat. Nous condamnons tous ici toutes les violences politiques et je veux associer à l'expression de notre dégoût face à ce qu'a subi Yannick Morez cet ignoble, passage à tabac avant-hier du neveu de Madame, Brigitte Macron. C'est aussi un acte inqualifiable et la justice doit être ferme dans un cas comme dans l'autre. Mais je vous demande précisément, Monsieur le Ministre de répondre aux interrogations de Yannick Morez. Nous lui devons cette clarté. Première question, pourquoi. Yannick Morel n'a-t-il pas fait l'objet d'une protection rapprochée de l'État depuis le mois de mars. 2ème question pourquoi avoir autoriser la manifestation aux qui date du 29 avril, un mois après l'incendie, véritable désaveu du maire qui avait pourtant demander son interdiction le 14 mai, Après de Callac après Saint-Brévin et avant d'autres drames. Allez-vous enfin interdire ce type de manifestation qui sont d'évidence d'appel à la haine de la part de l'extrême droite. Pour vous répondre. La parole est aux milices de air. Cohésion des territoires. D'abord. Vous me permettrez en saluant Yannick Morez de me réjouir de l'image que vient donner le Sénat. Puisqu'aucun membre des rester assis au moment de l'hommage qui lui a été rendu alors que nous avons assisté hier. Alors que nous avons assisté hier à l'Assemblée nationale a une scène où une partie de l'hémicycle ne s'est pas levé et je pense que ça témoigne précisément. Et je pense que ça j'aimerais. Prétendent défendre la liberté d'expression en empêchant quelqu'un de s'exprimer. Toujours quelque chose qui m'a semblé bizarre je commence ce propos en saluant le fait que tous les élus sur tous les bancs ici se lève alors qu'hier. Le Rassemblement national a refusé de se joindre à l'hommage. Et. Vous prétexté que compte tenu de la formulation de la phrase ça engendrerait la moindre gêne. C'est un début de récupération que de laisser penser. Qu'il y aurait une façon qui seraient à géométrie variable de décrire les choses. Et je veux saluer. Les propos de Ronan Dantec qui, sans la moindre hésitation et avec le sens républicain qu'on lui connaît. On a profité aussi pour rappeler les faits inacceptables subies par le petit neveu du président de la République dans un continuum de violence qui de cette manière-là se retrouvent. Mesdames et messieurs, vous avez ce matin. Reçu Yannick Morez dans le cadre d'une mission plus large portée par le sénateur d'Arnaud par l'avenir de la commune. Nous allons avoir trois, quatre, cinq questions qui seront autant d'occasions de de vous répondre dans les minutes qui viennent. Et je me réjouis que le Sénat, au travers de cet exemple. D'un acte de courage d'intimidation et d'un niveau de violence qui a été franchi et qui a atteint des paliers inacceptable essaye de faire la lumière. Ce que je souhaite dans le même temps, y compris compte tenu des retours que nous avons c'est que vous en profitiez peut-être pour demander. Aux forces de l'ordre à ceux qui travaillent au sein de Loire-Atlantique qu'elle a été leur version de leur côté les retours qu'ils ont eu dans les éléments qui nous sont données, il y a eu des patrouilles de police plusieurs nuits dans la foulée immédiate du 22 mars. Je vous dis ce que je sais, il y a eu des propositions qui ont été faites auprès d'Yannick Morez pour faire en sorte qu'il puisse bénéficier d'un accompagnement et des tentatives de prise de contact de la part de la préfecture ou de la sous- préfecture y compris dans la lecture de ce qui a été l'audition ce matin qui a manifestement sur l'absence de réunions publiques sur des manifestations qui se sont tenues des zones donc il convient d'éclaircir ce que je pense c'est qu'une commission aussi importante que celle-là sur un sujet aussi sensible nécessite sans doute que vous y passer encore un peu plus de temps que ce que vous aviez pu imaginer. pu imaginer. Quelques secondes monsieur Dantec. Il vous reste quelques secondes. Si vous le souhaitez. Oui. Juste Monsieur le Ministre, je crois qu'il n'y aurait pas de honte à reconnaître que sur cette affaire. L'État n'a pas été à l'auteur. Ça faciliterait les choses. L'État L'État notre collègue Joël Guerriau. Pour le groupe les indépendants République et Territoires. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, en novembre 2022. Le Sénat à l'initiative de notre collègue Nathalie Delattre a voté une loi promulguée en janvier dernier permettant aux associations d'élus, de se constituer partie civile pour se tenir les élus ou leurs proches, victimes d'agressions. Ce texte ouvre aujourd'hui la possibilité à Yannick Morez maire de Saint-Brévin d'être défendu par l'Association des maires de France. J'ai invité Yannick Morez aux tribunes et je suis très heureux de l'hommage que vous venez de lui rendre. En avril, j'ai animé en sa présence. Une réunion avec plus de 50 élus de Loire-Atlantique sur ce sujet. Tous ont témoigné d'incivilités et d'agressions dont ils font l'objet, il ressortait un profond mal-être et de la colère car les élus portent plainte. Mais bien souvent, rien ne change. Trop de plaintes sont classées sans suite et les auteurs recommence de plus belle. À titre d'exemple, le maire de Saint Père Henri commune voisine de Saint Brévin est agressé par le même individu depuis plus de trois ans. Hier, Jean-Baptiste Trogneux a été victime d'une agression odieuse uniquement parce qu'il est le petit neveu du président de la République. Ces agressions prennent aujourd'hui des formes multiples, certains se cachent derrière l'anonymat des réseaux sociaux pour harceler menacer insulter toute autorité publique et leurs familles. D'autres se rendent coupables de violences physiques. L'ensemble est favorisé par des discours haineux de certains responsables politiques on ne peut pas appeler à la violence et s'en laver les mains. Il faut que la justice passe avec fermeté. Il s'agit avant tout de dissuader en amont en sanctionnant des coupables par des mesures plus qu'aurait coercitive. Monsieur le Ministre, comment assurer à nos élus à leurs familles que la nation et l'État se tiennent à leurs côtés et que ces actes ne restent pas impunis. Pour vous répondre. La parole est au ministre de la cohésion des territoires, monsieur Christophe Béchu. Monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs. Je n'aurai aucune difficulté quand tu nous irons au terme de l'ensemble de la lumière qui est nécessaire sur. Ce qui s'est fait à Brévin à partager avec vous et le constat et la reconnaissance des dysfonctionnements, s'il y en a eu et je veux dire à Yannick Morez en le regardant. Que son exemple à beaucoup d'égards, ils nous oblige. Ce qui suppose de mesurer qui à la fois les actes pour lesquels des élus peu viande cause parce que ça correspond leur décision et d'autre dans lequel il s'agit d'aller partager une responsabilité nationale. Il y a un an, j'étais maire. Comme beaucoup ici. Les intimidations. Les invectives, les insultes, les trucs dans les réseaux sociaux les commentaires. Haineux. Les affiches, les tracts anonymes je connais. Beaucoup d'entre nous connaissent l'année dernière, ces 2265 atteinte à des élus. 32% de plus qu'en 2021. En face. Compte tenu à la fois du durcissement des textes 945 sanction pénale. Quand on a été capable de retrouver les auteurs, l'enjeu c'est de franchir de nouveaux paliers, Monsieur le Sénateur Guerriau d'abord pas seulement analyser comme le dit le président Kader mais faire un centre de coordination de la lutte contre les élus. Comment la justice. Comment la gendarmerie et la police sont en capacité les partager des informations par rapport aux menaces qui visent les élus et comment on est capable d'y répondre y compris en systématisant. Le suivi de la protection et de l'accompagnement des élus 2ème chose. Nous avons, vous avez parlementaire à une très large majorité considéré que le port de l'uniforme. Devait être une circonstance aggravante. Parce que quand on s'on prend un pompier, un gendarme ou un policier derrière l'uniforme c'est aux valeurs de la République qu'on s'attaque. Est ce que l'écharpe tricolore n'est pas à bien des égards. Une forme d'uniformes républicain qui mériteraient la même reconnaissance des circonstances aggravantes. Et ce que nous ne pourrions pas là aussi. Considérer que ce n'est pas seulement la personne du maire qui est visée mais sa fonction et à travers elle, ce qui lui ont été donné mandat c'est-à-dire la République et la démocratie. Merci Monsieur le Ministre. Dans le cas de Yannick Morez c'est l'accumulation de faits avant même qu'il y ait une réaction qui pose problème. Il aurait fallu très rapidement réagir. C'est avant tout le très classique qu'il s'agit de et pour cela, hé bien il faut absolument que nos coupables les coupables des faits hé bien et peur de notre justice. Merci la parole est à d'autres collègues Catherine Belghiti pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le garde des Sceaux. La démission de Yannick Morez maire de Saint-Brévin-les-Pins. Le 9 mai dernier a suscité indignation générale et un tollé médiatique sans précédent intimidé depuis des mois, abandonné par un appareil étatique restés sourds à ses avertissements. Celui-ci a finalement rendu son écharpe suite à l'incendie criminel de son logement familial dans la nuit du 22 mars dernier. Ce drame républicain est malheureusement loin d'être isolé. En effet, depuis le décès tragique du maire de signes en 2019 les agressions envers les élus de la République se sont multipliés, vous le disiez tout à l'heure Monsieur le Ministre, 2265 plaintes et signalements en 2022 soit une hausse de 32% en un an. Pire encore, selon le président de l'AMF David Linares le seuil fatidique des 1000 maire démissionnaire depuis les municipales de 2020 a été franchie, nous en sommes aujourd'hui à 1293. Démission. J'avais déjà eu l'occasion d'alerter le gouvernement sur la recrudescence des agressions envers les élus le 13 avril dernier. Madame la Ministre forme avait alors annoncé la création prochaine d'un centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus. Mais nous savons tous ce qui se passe sur le terrain. Un mois plus tard, aucune réponse pénale adaptée ne semble à l'ordre du jour et une certaine impunité règne pour les auteurs de ces agressions, à l'initiative du Sénat la loi du 24 janvier 2023, permet aux associations d'élus, de se constituer partie civile pour soutenir au pénal un élu victimes d'agressions. les sanctions ne sont pas à la hauteur. Monsieur le Ministre, combien de démissions supplémentaires faudra-t-il pour intensifier la répression envers les auteurs de ces attaques et préserver ainsi le pacte républicain. Pour vous répondre. La parole est à la ministre. Délégué en charge des collectivités territoriales. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs. Les sénateurs, madame la sénatrice Belghiti. Je voudrais tout d'abord évidemment me m'associer. À vos mots. Pour dire à quel point ces violences sont inacceptables, je veux redire à monsieur le maire. Tout mon soutien. Toute notre solidarité au nom de la Première ministre, au nom de Christophe Béchu au nom de Gérald Darmanin au nom de tout le gouvernement. Dans notre République cette inacceptable. Nous devons briser la spirale de la violence faite aux élus. On ne laissera rien passer cette violence. Est d'autant plus inacceptable que j'étais maire moi-même jusqu'au 7 juillet dernier et qu'on sait à quel point les maires et que vous représentez tous ici en fait sont les garants de la sécurité sur leur commune. De la protection de l'environnement de l'action sociale sur leur commune, ils sont dans l'intérêt général. On sait à quel point ils sont dans le don de soi. Cependant, je ne peux pas ne pas rappeler très brièvement à quel point nous sommes dans l'action, vous l'avez dit la sénatrice de Lattre. Ah permis par sa PPL. Le fait que les associations d'élus puissent se porter partie civile. Oui, c'est un élément. Oui, la loi qui a été porté en 2019 par notre collègue Sébastien Lecornu engagement et proximité vise à renforcer, comme l'a dit madame, la Première ministre, la protection des élus. Oui des circulaires, pas moins de trois qui ont été envoyées au parquet, demandant une réponse pénale ferme et rapide. est-ce que pour autant nous en restons là est-ce que pour autant nous voulons. Amplifier ce qui est fait, ce que nous voulons aller plus loin. La réponse est oui et là je m'adresse à vous monsieur le sénateur, qui n'avait cité que ce centre de lutte que ce centre d'analyse que j'ai cité effectivement dans un de mes propos, mais ce n'est pas que cela. Nous sommes aussi là pour d'abord et avant tout protéger les élus. Donc nous allons amplifier ce que nous faisons et j'aurai le plaisir de l'annoncer ce soir après avoir rencontré Monsieur le maire de Saint-Brévin aux côtés de madame, la Première ministre parce que l'action vous l'avez tous chevillée au corps, nous aussi, au gouvernement, nous l'avons chevillée au corps. L'action et donc ce soir. Je dévoilerai ce que nous allons faire à court terme là maintenant pour protéger nos élus, mais aussi je vous expliquerai pourquoi. Comprendre est important. Pourquoi ce centre de lutte est important. Pourquoi le choc civique est important et nous apporterons aussi madame la sénatrice, une heure. France-judiciaire, je vous remercie. Madame la Ministre, ce qui arrive à Monsieur Morel n'est pas isolée hein. Je crois que tout ce qui arrive, renvoie à l'incapacité chronique de réaffirmer l'autorité de l'État. L'urgence est là sans mesures répressives appropriées le mandat municipal est menacée et sans les maires, c'est la République elle-même qui menace ruine. Merci. La parole est à. Notre collègue Françoise Gatel pour le groupe de l'Union centriste. Merci, monsieur le Président les difficultés, les démissions s'enchaînent, et s'graines comme les questions aujourd'hui. Parce qu'il ne savait pas que ce serait ardue très difficile voire risqué. Beaucoup de citoyens se sont engagés juste pour servir. Hommes et femmes de devoir plutôt que de pouvoir les maires sont trop souvent contraints empêcher démunis submergé de normes et d'injonction. Mais il reste responsable de tous les voici aujourd'hui avec leurs familles confrontées au délitement et à la violence de la société qui les prend pour cible de la mort du maire de signes en 2019 à la démission si symbolique de monsieur le maire de Saint-Brévin que je salue avec beaucoup de respect. Démission et difficultés s'enchaînent, certes, des dispositions ont été votées mise en oeuvre, il faut l'Atmen car nous connaissons les remettre éduquer, protéger sanctionné et surtout prévenir et empêcher ceci suppose que le couple mère préfet que nous avons tant célébrer pendant la crise du Covid soit fort et puissant partout dans tous les territoires et auprès de tous les élus, a fortiori quand l'État charge amer d'exécuter une mission en son nom, madame la Ministre, Monsieur le mini je ne sais pas qui me répondra. Écoute émotions, nous le faisons tous. Je sais que ça n'est pas simplement votre attitude mais cela ne suffit pas quand ta mère doit détourné le regard devant ses agresseurs, il nous l'a dit ce matin quand ta mère et condamné à quitter la commune pour laquelle il s'est engagé et a changé de vie. L'heure est vraiment la détermination et à l'action. La démission du maire de Saint-Brévin. La démission des maires nous oblige Madame la Ministre quelles sont les intentions du gouvernement avant que vous voulez préciser à la télévision serait ravi de les avoir ici au Parlement. La parole est La parole est à la ministre. Délégué chargé des collectivités territoriales. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Gatel donc. Vous redire et le redire à monsieur le maire, il a tous les maires qui font l'objet de violences faites aux élus ces dernières semaines mais j'ai envie de vous dire tout à fait en introduction. Que le diagnostic nous le partageons. Que c'est par l'écoute, c'est par la proximité c'est par le respect les ont des autres. C'est par la solidarité mais aussi c'est par l'action, je vous le redis, Monsieur le Sénateur, que l'on va pouvoir endiguer cette violence faite aux élus. Alors vous parlez de la Préfet maires on le connaît tous ici il est efficace, il est à l'action. Alors bien sûr nous allons écouter monsieur le maire et nous allons écouter je l'coûterait aux côtés de madame, la Première ministre. Les raisons qui lui font percevoir que effectivement les services de l'État n'ont pas été à la hauteur de vos attentes et on va vous écouter et ça dans l'esprit de ce qu'a dit Christophe Béchu tout à l'heure de toujours s'améliorer, oui on va s'améliorer, de ce que vous allez nous dire monsieur le maire et de votre perception de cette inaction perçue par vous, moi je veux pas rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, on a le sentiment d'avoir agi. Cependant, on est vraiment à l'écoute et avec une envie chevillée au corps d'avancer. Alors vous me demandez de dévoiler quelques actions seulement il s'agit ici. De vous le dire en 2 minutes, donc c'est un peu court, me semble-t-il mais je voudrais juste citer un point un point. Ça s'appelle l'alarme élu ces 3000 référents dans la gendarmerie et dans la police nationale qui seront dès le début de la semaine prochaine, investi de une extrême proximité ce sera des référents violences aux élus. Ça a été décidé par le début de la semaine par Gérald Darmanin. Et c'est ce qui va faire juste si vous voulez bien m'écouter une seconde c'est super important. J'ai plus que 10 secondes à l'armée, lu ça veut dire qu'il faut que vous invitiez les maires à donner leur numéro de téléphone au préfet, aux gendarmes ou à la police pour que quand ils appelleront. Écoutez moi, pour que. Pour que quand ils appelleront ils puissent bénéficier d'un traitement spécifique, messieurs et mesdames les sénateurs. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Merci à vous. La parole est à notre collègue Cécile Cukierman. Pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les élus, leurs familles sont de plus en plus confronté à des actes de violence. D'agression d'intimidation parce qu'ils agissent pour l'intérêt de leur population de leur collectivité et de leur territoire. Je veux au nom de mon groupe, leur apporter tout mon soutien et redire qu'aucune violence n'est acceptable. La violence n'est pas dans l'ADN de notre sensibilité politique. Nous serons toujours dans le camp de ceux qui la condamne. La démission de notre collègue maire de Saint-Brévin les Pins n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle fait suite aux intimidations et menaces répétées de l'extrême droite depuis plusieurs semaines. Elle s'ajoute aux plus de 4000 démissions d'élus municipaux depuis 2020, dont plus de 1200. La non action ainsi que la banalisation de cette violence, permettent aux auteurs d'agir sans limite. Cela met en danger les élus leur famille mais aussi notre démocratie notre République. Nous devons donc redonner du sens à l'engagement le sacraliser. Nous avons tous notre rôle à jouer en responsabilité. Les communes qu'elles soient rurales, urbaines ou d'outre-mer demeure le 1er lieu de vie et de solidarité. Cellule de base de la République, elles doivent retrouver toute leur place dans l'organisation démocratique de notre pays. C'est une urgence démocratique c'est une urgence pour la République. comment entendez-vous redonner du sens à l'engagement de ces milliers d'élus locaux qui, au quotidien, agissent pour l'intérêt général et l'intérêt de chacune et de chacun, comment entendez-vous éviter de tels dysfonctionnements à l'avenir.

D'abord. Vous l'avez dit. Au-delà de Saint Brévin c'est plus largement le sens de l'engagement municipal le sens de l'engagement de mer que nous devons. Et mal nommer les choses. C'est ajouter aux malheurs du monde. La démission du maire de Saint-Brévin a été poussé par des manifestants d'extrême droite et provoqué par un acte scandaleux visant sa famille et son intégrité physique. Mais les 1293 d'missions depuis 3 ans. Elles n'ont pas toutes la même cause. Certaines sont liées à des violences de tous origine parfois sans arrière-pensée politique. Il y a la bêtise à des conflits de voisinage et dans d'autres cas à des affaires internes aux équipes à des difficultés par rapport au poids des normes à la multiplicité des réunions, à des difficultés dans une intercommunalité entre mer. En nombre de démissions. À mi-mandat. Nous en sommes au même nombre en ce qui concerne les mères. 1400 sur les 3 premières années du mandat 2014 2020. 1293. Quand on s'arrête au mois de mars. Sur les 3 premières années avec la parenthèse Covid qui bouleverse sans doute une partie de l'analyse puisque certains mandats ont commencé avec du retard. Je me réjouis de l'initiative transpartisane de l'avenir de la commune et je serais heureux d'être auditionné comme c'est prévu pour vous préciser ce à quoi nous pensons le sujet du statut de l'élu. La question du nombre de réunions et même je vais vous dire parce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez. Le statut du secrétaire de mairie du collaborateur qui permet de soulager de manière concrète le maire. Voilà une oeuvre utile pour faire en sorte d'avancer et de regarder comment on peut de manière intelligente, faire en sorte de limiter une part de la charge mentale qui accompagne la fonction municipale et puis collectivement. Telle que vous venez de le faire refuser toutes les violences. Refuser toutes les excuses à ceux qui décide du. Je lisais, autre chose que la démocratie pour remettre en cause des démissions, c'est le bon moyen parce que ça commence avec le coup d'école qui se justifie avec le courrier anonyme parce que le terrain est pas constructible, et ça se poursuit après par un changement de nature dans les actes, c'est au 1er signe que nous devons faire rempart collectivement pour protéger les élus. Je sais à quel point le Sénat dans sa plus la réalité. Est aux côtés des élus et se tient précisément pour faire en sorte de les préserver. La parole est à notre collègue Dominique Théophile pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes. Et indépendants. Vous avez la parole, mon cher collègue. chers collègues, mes chers collègues. Je salue bien sûr la présence du maire Yannick mauvaise et m'associe avec le groupe RDPI à l'hommage qui vient d'être rendu. Nous devons condamner toutes les formes de violence. Madame la Ministre, dimanche en Guadeloupe. Une mère de famille est mort au volant de sa voiture et la hausse. Une balle dans la tête. Mercredi, ce sont de jeunes hommes de 18 et 22 ans qui ont trouvé la mort au Lamentin et aux Abymes en Guadeloupe eux aussi par arme à feu. Ces drames, ce sont les derniers en date d'une liste qui ne cesse de s'allonger. Depuis le début de l'année une quarantaine de personnes ont ainsi. Été blessés ou tués par balle dans notre archipel sans qu'il ne soit permis d'espérer un retour au calme. Cette violence. Nous ne la découvrons pas. Depuis quelques années elle explose en Guadeloupe et en Martinique elle s'accompagne d'un phénomène de gangs. Et se nourrit du trafic d'armes à feu qui déséquilibre la caraïbe et qui ensanglantent Haïti. Les pouvoirs publics ont pris la mesure de ce phénomène et il me faut saluer le travail exceptionnel des forces de l'ordre et des fonctionnaires de justice. Il y a quelques mois. C'est une vaste opération menée sous l'égide d'Interpol, qui a ainsi permis la saisie d'armes et de munitions. Cette réponse. Pourtant, n'est pas suffisante. Elle le sera quand cesserons c'est des dresser drame qui endeuille chaque semaine des familles. Madame la Ministre quelles réponses supplémentaires. Entendez-vous apporter pour enrayer ce cycle de violence. Comment mieux lutter contre un trafic d'armes qui dépasse de loin nos frontières, les collectivités locales, la société civile et les familles sont engagés dans ce combat au quotidien. Elles attendent de l'État une réponse forte et déterminée ne pourront pas tenir les armes si aucune comme un achat dans un commerce. Pour vous répondre. La parole est à la ministre. Déléguée en charge des collectivités territoriales. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Théophile. Vous avez raison. La Guadeloupe et la Martinique connaissent depuis quelques années, une hausse des violences avec arme et les homicides. L'utilisa Sion d'armes à feu est en constante augmentation et tend à se banaliser. Avec une utilisation régulière par des primo-délinquants dans le but de se protéger en Guadeloupe de 130 armes ont ainsi été saisis dans ce cadre en 2022. Ce qui démontre la banalisation du transport et du port d'armes sur le territoire. Alors des actions de prévention d'abord campagne de communication et diffusion de messages télévisuels sur les chaînes locales et sur les réseaux sociaux, financés par le fond le FIPD mais vous le savez réunions régulières de concertation avec la société civile afin de développer de plus en plus de bonnes pratiques mais aussi la multiplication des opérations de contrôle mené à l'appui d'arrêtés préfectoraux spécifique interdisant la vente, la détention et le transport d'arme de catégorie C 3 aider sur le territoire de ces 2 départements. Ensuite, le développement, le développement des moyens d'enquête judiciaire notamment d'enquêteurs spécialisés. Spécialisé cyber chargée d'enquêter sur la vente et l'achat d'armes par Internet en 2022. Un enquêteur nouvelles technologies de la gendarmerie ainsi contribuer à l'identification de plusieurs trafiquants et au démantèlement d'un atelier de transformation de pistolet d'alarme en armes létales situé sur la commune du Robert. La coopération avec les États voisins relance des échanges avec. Lucie, dans le cas de la commission mixte. Renforcement de la coopération avec la maréchaussée de Saint-Martin. Tout ça vous le savez, mais il faut poursuivre renforcer soyez convaincu monsieur le sénateur de l'engagement total. Du ministère de l'Intérieur pour et de l'outre-mer pour continuer la lutte contre les trafics à Marseille, pas seulement en Guadeloupe et à la Martinique, merci. La parole est à notre collègue Arnaud Bazin pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, madame, la Première ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. On avait bien compris à l'été 2021 s'étaient juré le quoi qu'il en coûte c'est fini. Pour la loi de finances 2023 le montrant avaient un peu changé. C'était chaque euro compte. Et en même temps depuis quelques semaines, le président de la République et le gouvernement rivalisent d'annonces de dépenses nouvelles supplémentaires par centaines de millions, voire par milliards d'euros, 2 milliards d'euros pour le plan vélo de milliards d'euros de baisse pour l'impôt des classes moyennes. Un milliard d'euros pour les lycées professionnels. Cela peut représenter 18 milliards d'euros en cumulé d'ici la fin du quinquennat. Dans le même temps les intérêts de la dette cette année vont augmenter de 12 milliards d'euros. Bientôt le service de la dette sera le 1er budget de l'État et l'impôt sur le revenu des Français n'y suffira même plus. Dans le même temps les prévisions économiques du gouvernement. Nous les avions jugé optimiste en examinant la loi de finances 1% de croissance. Ce n'est pas ce que nous observeront le P.. Le FMI avait dit 0 6 % c'est sensiblement, ce qui se confirme dans les premiers chiffres que nous avons. Alors dans ce contexte. Incertain pour ne pas dire inquiétant des finances publiques. Quand cette baisse d'impôt en faveur des classes moyennes pourra-t-elle avoir lieu. Pour vous répondre. La parole est aux ministres. Délégué en charge des comptes publics. Monsieur Attal. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur. Bazin vous aborder des sujets que nous avons longuement évoqué ici même lors du débat d'orientation des finances publiques. Il y a quelques jours au cours d'une soirée avec le rapporteur général Husson. Le président rénal et beaucoup d'entre vous. D'abord la l'annonce du président de la République sur la baisse d'impôts pour les classes moyennes. Je veux rappeler qu'elle s'inscrit dans une politique résolue de renforcement du pouvoir d'achat des Français qui travaillent, qui nous a amenés à la suppression compenser de la taxe d'habitation. Ah la redevance télé qui a été supprimé à la baisse de l'impôt sur le revenu pour les 2 premières tranches à la défiscalisation des heures supplémentaires et à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Cette politique, elle a un sens, c'est redonner de l'oxygène à tous ces Français qui se lève le matin qui travaillent et qui ont parfois le sentiment qu'ils financent avec leurs impôts. Un modèle qui permet à certains de ne pas travailler ou des services publics qui se dégradent, ce qui nécessite pour nous évidemment de leur redonner du pouvoir d'achat et d'agir sur la qualité de la dépense publique. Pourquoi est-ce que cette politique et n'est pas contradictoire avec le rétablissement des finances publiques parce que quand vous prenez des décisions de diminution de fiscalité qui ont un impact positif sur l'activité économique dans notre pays. Vous avez des recettes supplémentaires. On a passé l'impôt sur les sociétés de 33% à 25% on collecte plus d'impôt sur les sociétés depuis que le taux est à 25% qui à l'époque où il était à 33%. Les décisions qui permettent de renforcer l'emploi dans notre pays, de rendre plus attractif l'emploi et l'activité économique sont aussi bonne pour les finances publiques. Pour le reste j'ai annoncé et j'ai présenté lors du débat d'orientation des finances publiques, la trajectoire budgétaire pour les 5 années à venir, issus du programme de stabilité. Nous allons ramener notre déficit à 2,7% en 2027. Nous avons tenu ces dernières années tous les objectifs de déficit que nous avions fixé il a diminué chaque année et s'agissant du cadrage macroéconomique et des doutes sur les prévisions de croissance. Je veux rappeler qu'ici même il y a un an j'entendais certains douter d'une croissance à 2,5% en 2022, nous l'avons dépassé et qu'à l'Automne dernier certains remettait en cause le fait que nous aurions une croissance positive en 2023 et que les prévisionnistes sont en train progressivement de s'aligner sur notre prévision à 1% de croissance pour cette année 2023, le FMI que vous avez à 08. L'OCDE est à 0 7 oui, nous avons une économie qui résiste parce que nous avons des entreprises qui embauchent et qui investissent, c'est bon pour le pays, c'est bon pour l'emploi et c'est même bon pour les finances publiques. Je vous remercie.

quand la trajectoire des finances publiques le permettra, à travers les documents budgétaires que vous avez rappelé. Paraîtrait raisonnable. Disons moins déraisonnable d'envisager cette baisse à l'échéance du présent du pressé En conséquence, les Français auront bien compris que la situation des classes moyennes s'améliorera quand Emmanuel Macron ne sera plus président de la République. La parole est à neutre. Collègue Marie-Arlette Carlotti pour le groupe socialiste écologiste. Merci Merci monsieur le président. À Marseille la pègre tu es le tu sur fond de vendetta entre bandes rivales régnant sur les trafics de stupéfiants depuis le début de l'année. Marseille vit au rythme d'un assassinat par semaine et les réseaux en plus que jamais la mainmise sur le quotidien des habitants car les gangs ne se tue plus entre eux ils ont font de plus en plus de victimes collatérales des enfants de 15 ans, assassiné une femme tuée au volant de sa voiture, lors d'un échange de tirs. Un homme atteint d'une balle perdue alors qu'il jouait au bas aux cartes, au bar du coin. Un jeune tué aux jambes tout touché aux jambes par une rafale tirée à travers le sa porte d'entrée comme ça. Fusillade à l'aveugle, séquestration. Mortel diffusé sur les réseaux sociaux, les trafiquants imposent leur terreur avec mon collègue Jérôme Durain. Nous sommes allés à la rencontre des victimes de leur famille, de la population qui se sent impuissante vulnérable abandonnée, impuissante parce que assignée à résidence parce qu'elles n'ont plus les moyens de quitter leur cité HLM des quartiers qui sont mal irriguées en transports en commun des déserts médicaux et des écoles insalubre que le maire de Marseille à la volonté de réhabiliter déjà déjà ils avaient le sentiment que la République les avait abandonnés. Mais désormais, ils savent que, chaque jour ils risquent leur vie car il ne faut pas se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. La police pilonne les points de deal fait des records de de prise de shit c'est bien mais à l'évidence, ça ne marche pas. Vous avez déployé des moyens importants notamment sur Marseille, ça ne suffit pas. C'est donc sur votre doctrine que je vous interroge, est-ce que vous croyez par exemple que c'était vraiment le moment d'affaiblir la police judiciaire alors que leur objectif c'est justement de démanteler les réseaux. Oui, la guerre des gangs. Nous l'avons entendu sur ce ce réparties partout dans le pays et nous aurions tort de penser que cette situation n'est propre qu'à Marseille nous ici, nous soutenons les forces de l'ordre. Nous respectons la police mais quand les choses ne fonctionnent pas. C'est au ministre à revoir sa copie. Alors aujourd'hui Madame la Ministre au-delà de Marseille. C'est pour toutes les villes de France que nous nous indignons et que nous vous demandons, ce que vous comptez faire. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Carlotti oui nous partageons ce constat inacceptable. En fait depuis le début de l'année ce sont 17 personnes qui ont été tués dans le cap domicile liés au trafic de supprimer de stupéfiants. Et je voudrais ici au nom de Gérald Darmanin de madame, la Première ministre et de tout le gouvernement. Avoir un mot pour leurs familles et leurs proches endeuillés. Mais face à cette situation intolérable là où nous divergeons c'est que le ministère de l'intérieur des Outre-mer est pleinement mobilisés d'ores et déjà c'est pas ce que nous comptons faire c'est ce que nous faisons et si vous me le permettez, je vais le rappeler entre 2021 2022 c'est 300 policiers qui ont été dépêchés en renfort et contrairement à ce que vous disiez en début d'année c'est 10 nouveaux policiers qui sont venus renforcer la police, la police judiciaire et qui permettent de créer un groupe supplémentaire pour l'Office anti-stupéfiants ces 3 compagnies de CRS qui ont également été affectées en permanence à Marseille, soit un total de plus de 140 policiers, c'est 30 jeunes policiers en sortie d'école, qui ont été affectés à Marseille depuis le 2 mai, madame la sénatrice 11 nouveaux policiers arriveront à la police judiciaire d'ici septembre pour renforcer la brigade de recherche et d'intervention 90 postes qui ont été ouverts. Rien que sur Marseille. Dans le cas du prochain mouvement de mutation et qui arriveront en septembre prochain. Enfin, grâce à la Lopmi que vous avez voté en ce début d'année une nouvelle compagnie de type CRS. Numéro 8 sera implanté à Marseille et même d'ici la fin de l'année 2023. Cette politique montre des effets concrets d'ores et déjà madame la sénatrice bien sûr insuffisant mais il me faut le rappeler, de janvier à mars 2023, ce sont 362 opération visant des points de deal

De nous interroger mais entendait les réponses que nous apportons. D'ores et déjà je vous remercie. Merci la parole est à notre collègue Max Brisson. Pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale. Après un long silence vont entrer en scène était particulièrement attendu. On vous annonce. Loin de répondre au besoin de réforme de l'école fut pour fuir plus polémique que saluer. Elles ont cependant ouvert de nouveau débat sur la laïcité et la mixité sociale. J'ai donc 3 questions à vous poser. À l'aune de la composition du nouveau conseil des sages de la laïcité. Entendez-vous redéfinir ce principe fondamental d'autres républiques qui prévaut jusqu'à présent à l'école publique alors que le chef de l'État vous invite à ne pas réveiller de vieux conflit pourrait vous présenter un jour votre plan sur la mixité sociale à l'école finalement, Monsieur le Ministre, avez-vous la confiance du président de la République pour réformer et diriger l'éducation nationale. Je vous répondent. La parole est. Ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, monsieur Pap Ndiaye. Brisson. 3 questions ou plutôt. Ou plutôt de auxquelles je vais répondre successivement la première. Porte sur les questions de laïcité. J'ai eu l'occasion déjà de m'exprimer devant vous pour. Indiquer que d'une part la laïcité doit être observé de manière ferme et strict, nous devons respecter strictement la loi de 2004 qui est notre boussole en la matière. Être ferme à l'égard de celles et ceux qui contreviennent au principe de laïcité et depuis l'Automne il y a eu des conseils de discipline, il y a eu des sanctions qui ont été prononcées. Mais j'ai également eu l'occasion de dire que la laïcité, c'est aussi une pédagogie la laïcité ne doit pas seulement être crainte elle doit être aimé. C'est ce que disaient les républicains à la fin du XIXe siècle, la République ne doit pas être crainte seulement, elle doit être aimé. Nous devons donc développer une pédagogie de la laïcité, c'est très important pour convaincre et ne pas simplement faire respecter au sens strict du terme. Nous avons pour cela un conseil des sages qui orientent l'action du ministre fournit des éléments intellectuels des éléments de doctrine et nous avons aussi en parallèle une administration avec plus de 600 personnes dans les équipes valeurs de la République qui travaille à faire respecter la laïcité sur le terrain de façon ferme avec discernement mais de manière très ferme. En ce qui concerne votre 2ème question je vais dévoiler ce soir puisque nous allons signer un accord avec le secrétariat général de l'enseignement catholique pour ce qui concerne le privé et une batterie de mesures en ce qui concerne le public de nature à favoriser la mixité car la mixité, c'est bon pour le climat scolaire, c'est bon pour le climat social c'est bon pour le niveau des élèves. C'est bon aussi pour la laïcité. Monsieur le Ministre, acteur. Le président de la République face caméra multiplie depuis un an, les annonces sur l'organisation scolaire et son évolution. Acte de seule et en militant pour enfin exister vous concentrer sur 2 sujets une laïcité à géométrie variable qui conduit au torpillage du conseil des sages et qui laisse sans directives proviseurs et professeurs, puis en 6 moulage éculés de l'enseignement privé qui serait vieux fantasme de gauche la source des défaillances de l'enseignement public. Acte 3, le président République vous rappelle à l'ordre et vos plans sont rangés au placard. Le problème est qu'à force de tirer à Hue et à Dia. La rue de Grenelle et l'Élysée passe à côté de l'essentiel. La réforme de service public à bout de souffle. Cessez donc de jouer avec l'Élysée ce bien mauvais Vaudeville. Monsieur le Ministre,

Madame, la Première ministre, mesdames, messieurs les Ministres, chers collègues, ma question concerne les mineurs non accompagnés. Une question qui n'est pas nouvelle et qui demande une réponse en fait interministériel parce qu'elle peut aussi bien avoir une réponse sur le plan du ministère de l'Intérieur pour les flux migratoires que sur la justice avec l'évaluation de la minorité. Que sur la solidarité que sur la protection de l'enfance que sur l'éducation même le travail quand tu nous avons des chefs d'entreprise qui demande à ce que on puisse maintenir. Des jeunes sur notre territoire pour assurer soit des apprentissages ou du travail dans nos entreprises artisanales. Donc c'est vraiment un ensemble de réponse qui est attendue et aujourd'hui le cri d'alarme est lancé par le président de l'association des départements de France, François Sauvadet, qui dit que la situation est alarmante et il a raison. La situation est alarmante. 5000 mineurs non accompagnés qui sont arrivés depuis le début de l'année et notamment 2000 dans les Alpes Maritimes et je voudrais rappeler le chiffre entre 2021 et 2022 c'était 900 mineurs non accompagnés en plus dans le seul département des Alpes-Maritimes et la situation est vraiment catastrophique. Nous devons agir et je voudrais vous poser tout simplement cette question, va-t-on parler dans la loi immigration de cette question des mineurs non accompagnés. Il n'y a rien à ce jour dans cette loi concernant les jeunes alors que nous devons et les accompagner avec humanité, mais aussi avec responsabilité et faire en sorte que les choses soient acceptables aussi pour l'ensemble de la population, nous devons aussi. Penser à ce que nous avons voté dans la loi taquet, c'est-à-dire du 7 février 2022, nous avions 3 articles qui étaient concernés par les mineurs non accompagnés aujourd'hui rien n'est possible puisque ça ne s'est. Ce n'est pas passé au Conseil d'État. La 3ème question c'est, comment comptez-vous faire pour aider financièrement les conseils départementaux qui sont à bout de souffle aujourd'hui et les moyens financiers ont diminué ces dernières années. Je vous remercie. Pour vous répondre. La parole est à la ministre. Déléguée. En charge des collectivités territoriales. Merci monsieur le président. Mesdames, vous avez les sénateurs, madame la sénatrice Doineau. Avec le ministre de l'Intérieur, des Outre-mer, Gérald Darmanin, nous sommes pleinement mobilisés sur cette question et vous le savez des mineurs étrangers non accompagnés. Qui est à la fois complexe mais cruciale pour nos territoires et nos départements. Et pour eux bien sûr madame. C'est une question particulièrement actuel puisqu'en 2022, quelques chiffres, ils étaient 14.782 cas ils était 11.315 et les remontées des départements qui ont la charge comme vous l'avez indiqué, de l'accueil de ces jeunes montrent une augmentation prévisible de ces chiffres cette préoccupation, nous la partageons. C'est pour cela que la mission nationale des mineurs non accompagnés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la Jeunesse et pleinement mobilisés et à l'écoute des remontées des départements. C'est encore pour cela que je suis personnellement en contact régulier avec le président des départements de France, cher François Sauvadet. C'est pour cela, évidemment qui a été organisée avant-Vendôme la semaine dernière, une rencontre avec le ministre de l'Intérieur. La secrétaire d'État à l'enfance et qu'ils ont reçu ensemble les élus, les représentants du département des Alpes-Maritimes tout particulièrement exposés dans ce contexte, nous allons ainsi. Apporter des réponses concrètes à la situation de tension que vous avez décrite et que nous partageons et que connaît ce département en particulier mais comme vous l'avez dit, que connaissent aussi autres. Ce département soutien aux équipes départementales, en charge de l'évaluation, recherche de la mise en oeuvre des solidarités inter-départemental. Suspension de la clé de répartition concours exceptionnel de l'État. Toutes ces pistes sont à l'étude actuellement pour améliorer encore notre dispositif en lien avec les collectivités et tout particulièrement avec l'association des départements de France, le soutien de l'État au département dans cette mission très sensible. très sensible. Et Total offrir assez mineurs la prise en charge nécessaires est indispensable comme vous l'avez indiqué comme nous devons préserver tout comme nous devons préserver les équilibres de notre République et des territoires également. Je vous remercie. Merci la parole est à notre. Collègue Philippe Dominati pour les républicains. Merci monsieur le président, madame la ministre, il y a quelques jours un quotidien a publié son enquête annuelle concernant l'inquiétude des Français vis-à-vis de leur liberté individuelle. 64% d'entre eux considèrent que les atteintes à la liberté individuelle, se sont aggravées, au cours de la dernière décennie. Ce chiffre est également répartis entre les électeurs de gauche. Plus de 70%. Les entreprises 78%. Évidemment. Les les autres. Catégories de Français. Les interdictions pleuvent. Elles sont quotidiennes, les collectivités territoriales il participe. Je n'ai pas le temps évidemment de les énumérer, mais ça va de la possibilité de se laver d'arroser de chasser de choisir son médecin, sa santé se faire vacciner ou pas se faire vacciner de choisir sa fin de vie. Pour autant, les Français sont les citoyens les plus prodigues vis à vis de du pays. Il paye la dette. Il paye les impôts les plus élevés des démocraties. Ils payent le plus grand nombre d'agents publics. Et l'État mord la main de ceux qui les nourrissent. Je suis un républicain. Je ne suis pas fan des monarchies parce que je suis toujours étonné de voir que des contribuables pas. Payer ou enrichir le Patrimoine de leur prince mais force est de constater. Que entre le millier d'anglais qui est au sacre de Charles III. Et la pauvreté. La solitude de notre président de la République sur les Champs Élysées entouré de 10 policiers pour un spectateur, je m'interroge. Ma question est de savoir. Madame, la Première ministre ou Madame la Ministre, quelles instructions vous donnez à votre administration pour avoir les précautions de ne plus enquiquiner les Français au nom des précautions élémentaires. Au nom de la frilosité de votre gouvernement. Pour vous répondre. La parole est à la ministre. Délégué chargé des collectivités territoriales. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, vous interroger le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald. Darmanin sur un récent. Monsieur le sénateur Dominati. Sur un récent sondage de l'IFOP. Personne bien entendu ne concerne 2 conteste le sérieux de l'institut IFOP. Mais nous ne perdons pas de vue qu'on parle ici d'une perception subjective d'un sentiment. Si on s'en tient la réalité des faits et du droit. Nous souhaitons insister sur le fait que nous sommes dans un état de droit et que l'action du gouvernement. Tout comme celui des forces de l'ordre et guidés par nos principes constitutionnels et nos règles juridiques que nous partageons tous la liberté d'expression. Et en son sein la liberté de manifestation sont des principes constitutionnels auxquels nous sommes tous attachés. Mais nous rappelons également que des restrictions aux libertés individuelles sont possibles dans notre État de droit sous condition bien évidemment. Ainsi, les restrictions à la liberté de manifester. Doivent être strictement proportionnées au motif d'intérêt général à défendre. Les restrictions à la liberté de manifester doivent aussi être motivé par un risque avéré. De troubles à l'ordre public. Alors vous le savez peut-être monsieur mais ça me semblait opportun de le rappeler. Je rappelle également que dans notre pays. Toute restriction aux libertés individuelles et soumis au strict contrôle d'un juge des arrêtés préfet. Toro d'interdiction de manifestations ont déjà été confirmée par le juge mais faut-il rappeler que d'autres arrêtés préfectoraux d'interdiction de manifestation ont aussi été annulé par la justice. Alors quelques exemples, un colloque de l'Action française autorisée par le tribunal administratif. Samedi 13 mai, alors que le préfet de police avait pris un arrêté d'interdiction. Une manifestation organisée par la même action française dimanche 14 mai qui a défilé en hommage à Jeanne d'Arc, la démonstration est ainsi faite que nos institutions fonctionnent et que l'état de droit. Et respecté. Je vous remercie. La parole est à madame la présidente Laurence Rossignol pour le groupe socialiste. Écologiste et républicain. Merci monsieur le président je vais changer de sujet, essayer d'offrir un petit moment de pause à Madame la Ministre fort qui l'a bien mérité. Alors en 40 ans, un quart des oiseaux, c'est-à-dire 800 millions d'oiseaux ont disparu en Europe. Non non non. Ne vous laissez pas aller ses plaisanteries faciles. Et cet effondrement est directement imputable aux pesticides et à l'agriculture intensive. Chaque année, 300.000 personnes dont 12.000 enfants meurent prématurément de la pollution de l'air en Europe. Le niveau des nappes phréatiques est dramatique. Et l'Europe du Sud brûle déjà alors que nous sommes loin de l'été encore. Et voilà que le président de la République. Annonce vouloir une pause. Dans la réglementation environnementale européenne. C'est consternant. Et c'est d'autant plus consternant que de directives majeurs sont actuellement en discussion. La directive concernant les pesticides et la directive concernant les produits chimiques et être au sein discussion le Green Deal avec la question du principe du pollueur-payeur. Et avec ses déclarations. Est ce que le président de la République ne rapprocherait pas en fait la France du côté obscur de la force, c'est-à-dire de ces pays qui font le choix de céder le dis aux lobbies économiques et qui font le choix du cynisme de d'efficacité économique immédiate au détriment de la santé des Européens. La France risque avec cette déclaration. Si c'était si elle était confirmée. De torpiller les efforts que l'Europe doit faire pour accélérer sa transition écologique. Alors nous sommes dans une course de vitesse aujourd'hui contre la destruction du vivant. Nous sommes dans des difficiles négociations dans l'Union européenne. Dans quel camp et la France qui faut-il croire. Et ce qu'il faut croire le ministre Béchu qui au 1er janvier nous souhaiter à tous une année d'accélération de la transition écologique ou est-ce qu'il faut croire le ministre-Lescure qu'il demande 50 postes de la transition écologique.

D'abord merci d'avoir. Fait écho à cette étude hier qui pointe. Cette disparition inquiétante. De la mortalité des des des oiseaux à l'échelle européenne et les causes qui sont avérés. Nous sommes à quelques jours. D'une séquence très importante à l'UNESCO de la négociation. D'un traité sur la fin de la pollution plastique qui va se tenir en France. Parce que le président de la République l'a souhaité. Je suis heureux que vous m'interrogiez sur ces propos qui ne doit pas être mal compris. D'abord dans quel cadre ça se passe dans le cas d'une conférence de presse, choisi par le président de la République à l'Élysée pour expliquer qu'il faut accélérer sur la réindustrialisation écologique du pays. Et ça commence par une diapos projetées qui est celle du GIEC pour expliquer ce qui se passe et pour dire que nous devons changer de braquet parce que pendant trop d'années, on a baissé nos émissions en 18 industrialisant et que l'écologie ce qui en parlent le plus sont pas nécessairement ceux qui ont fait le plus. Sous le quinquennat que vous avez ardemment soutenu la baisse des émissions était de 1% par an, elle a été doublé pendant le dernier quinquennat et l'ambition de la doubler à nouveau ce qui a été annoncé ce jour là, c'est que nous allons nous saisir d'un texte européen négocié par le président de la République le Net zéro pour faire en sorte de pouvoir attribuer des subventions aux projets qui correspondent à une excellence écologique, environnementale dans un cadre qui est celui de la planification écologique souhaitée par le Haut Conseil pour le climat, confiée à la Première ministre de manière à assurer la transversalité. Le sujet s'est vu le nombres de textes qui viennent d'être voté et ceux qui sont encore devant nous riche et sur. Dans quelle mesure nous faisons en sorte maintenant de mettre les financements. C'est la phrase du président de la République pour appliquer les dispositions qui ont été prises plutôt que d'ajouter des textes à des textes alors que nous en avons déjà beaucoup de vent nous un exemple euros 7. On a il y a quelques mois dit ensemble qu'il fallait qu'on aille vers la planification de la transition écologique des voitures avec l'électrification dans le même temps l'évolution de la norme ne doit pas concerner le moteur c'est la pause mais ce compte rentrer sur les autres éléments, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'expliquer qu'on doit intensifier notre action sur la base des textes existants, qui sont déjà nombreux, tout en continuant négocier de nouveaux mais en ajoutant pas chaque jour le texte qui vient remplacer le précédent. L'ambition est totale. La Poste n'est pas pour l'ambition. Monsieur le président, Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Madame la Ministre en juin 2022 la Commission européenne a publié une proposition de règlement intitulé Loi sur la restauration de la nature. Il s'agit de l'une des mises en application de la stratégie européenne du Pacte Vert dans ce contexte, la commission Environnement du Parlement européen qui examine au fond le projet de règlement doit entériner sa position le 15 juin prochain. Dans son article 10, la loi prévoit que les États membres de rang devront écoutez bien augmenter la quantité de bois mort debout et au sol la connectivité forestière. Les stocks de carbone organique dans les sols ainsi que la part de forêt d'âge différent avec une hausse de tous ces éléments qui devra être mesuré tous les 3 ans dans l'ensemble des États membres, à compter de 2030. Cet article contrevient donc complètement à la doctrine française de lutte contre les incendies de forêt que nous avons ici au Sénat renforcés et sécurisés avec l'adoption de la proposition de loi de nos collègues j'Embassy Act Anne-Catherine Loisier, Pascale Martin et Olivier Athmane visant à renforcer la provision la prévention pardon et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie et qui prévoit entre autres de gérer d'améliorer l'aménagement et la valorisation des forêts en appréhendant la défense contre les incendies, à l'échelle du massif de financer la reconstitution de forêt plus résiliente après l'incendie aussi Madame la Ministre concernant ce texte européen de restauration de la nature. Quelles sont les actions françaises entreprises pour faire reconnaître l'expertise et le particularisme français en matière de lutte contre les feux de forêt. Pour vous répondre. La parole est à la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Madame la sénatrice du Mont en fait le 4 avril, le Sénat a adopté et vous l'avez dit à l'unanimité. J'étais au banc. Une proportion une proposition de loi ambitieuse visant à renforcer les moyens de. Prévention et de lutte contre les incendies.

les incendies que nous avons connu l'été dernier qui frappe déjà les Pyrénées orientales, à l'heure où je vous parle nous rappelle l'urgence d'agir face à ces phénomènes amplifiée par le réchauffement climatique et je profite de votre question, pour rappeler l'engagement de nos sapeurs-pompiers. Professionnels ou volontaires, et je tiens à leur apporter à votre nom à tous, tout notre soutien concernant le sujet spécifique du bois mort, aucune règle européenne ne se pose de manière générale, sur une parcelle forestière à l'enlèvement de ce bois mort dans une logique de prévention des incendies. Tout particulièrement. Cet aspect revêt même un enjeu important dans la prévention des feux de forêt et dans la limite. De leur propagation, la réglementation dite Habitat appliquée par l'article L 401 tirer 1 du code de l'environnement empêche pour sa part la destruction de l'habitat d'une espèce protégée, ce point précis n'empêche pas l'enlèvement du bois mort sur une par alors en ce sens, la réglementation européenne actuelle et la réglementation dite habitat nous semble concilier le double enjeu de préservation des habitats et de la biodiversité. D'une part mais aussi de prévention et de lutte contre les incendies. Je vous remercie, je suis ouverte à tout échange sur ce sujet. Je vous recevrai bien volontiers sur ce sujet sur lequel on travaille déjà depuis plusieurs mois ensemble. Merci.

pour nos massifs forestiers et bien sûr la mission de nos soldats du feu. Merci. La parole est notre collègue Olivier et nos pour le groupe de l'Union centriste. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre de la ville et du logement. J'espère ne patron contrarier Madame la Ministre qui vient de s'exprimer précédemment. Elle concerne le fameux DPE. Je n'aime pas les acronymes mais il faut s'y faire DPE diagnostic de performance énergétique j'associe à ma question. Jean Michel Arnaud sénateur des Hautes-Alpes très investi sur cette question. Monsieur le Ministre. Je ne remets pas en cause la bonne intention originelle du DPE. Mais depuis, Bernard de Clervaux. Nous savons que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Peut être allez-vous nous convaincre mais nous voyons de nombreux inconvénients à cette. Mise en place précipitée du DPE je cite les délais très contraints. Pour la réalisation des travaux et donc le renchérissement des coûts. La question du deux poids deux mesures entre les petites surfaces et les grands logements son caractère uniforme jacobin verticale et descendant on a malheureusement l'habitude qui n'indique pas les variations qui ne tient pas en compte, qui n'intègre pas les variations climatiques et c'est un homme du Nord qui parle et enfin ses conséquences sur l'offre de logements. Combien de logements vont disparaître de l'offre de location au moment même où se profile une crise du logement sans précédent. Pour conclure, vous l'avez compris, pour nous le DPE comporte des germes de fracture sociale et territoriale et donc ma question est la suivante, comment voyez-vous la mise en oeuvre du DPE son calendrier et ses conséquences sur la crise du logement qui se profile. Je vous remercie. Pour vous répondre. La parole est aux délices délégué en charge du logement. Merce. Klein. Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Olivier Henno. Oui. Le le DPE est utile. Le député a été réformée pour être plus en phase avec la réalité de la qualité des logements et il y a effectivement une crise du logement. Mais cette crise du logement ne doit pas nous laisser entendre qu'on peut laisser vivre nos concitoyens dans des passoires thermiques le calendrier tel qu'il existe aujourd'hui, il concerne d'abord pour le 1er janvier 2025, les plus. Les passoires thermiques, les plus importantes à partir. Des des étiquettes et puis 2028 F et Les propriétaires bailleurs comme les propriétaires occupants sont accompagnés et connaissent cette évolution depuis de nombreuses années d'ailleurs, les propriétaires bailleurs continue à à percevoir un loyer et pour ma part et je crois que c'est notre. Position à tous, on ne peut pas laisser des habitants vivre avec des enfants dans des passoires thermiques dans le fait qu'elle il fait très chaud l'été très froid l'hiver, dans lequel il y a de la moisissure sur les fenêtre s'et c'est le sens de cette mesure, le gouvernement agit à travers la mise en place de France rénovent à travers la, la mise en place dès cette année des accompagnateurs rénovent à travers ma prime Rénov'qui se développe notamment MaPrimeRénov sérénité qui doit accompagner les plus fragiles à travers le le doublement du déficit foncier qui va permettre aux propriétaires d'ailleurs d'être encore mieux accompagner. Dans leurs travaux et donc toutes ces mesures mises Boutabout doivent permettent de tenir ce calendrier parce que ce calendrier, il est dans l'intérêt de ceux qui vivent dans les passoires thermiques, notamment les plus fragiles de nos concitoyens. Ensuite je n'ai pas un certain nombre de particularités qui doivent être regardées notamment dans les territoires de montagne ou dans un certain nombre de cas et c'est aussi pour ça qu'il faut travailler à la rénovation thermique de l'habitat l'habitat collectif, parce que bien évidemment, un propriétaire qui a son appartement classé G dans un immeuble dans lequel on aurait rien fait, hé bien se retrouver en situation d'impossibilité de faire et c'est l'obligation qui nous est donnée, c'est de mieux accompagner l'habitat collectif dans ces travaux de rénovation. Je vous remercie.

perplexité lors de la mise en oeuvre et abandon en race campagne à l'approche du mur de la réalité. Je vous remercie. Nos prochaines questions d'actualité auront lieu le mercredi 24 mai à 15h je vais suspendre la séance elle sera reprise à 16h 30 pour l'examen de la proposition de résolution en application de l'article 34, tiré à la Constitution relative à la reconnaissance du génocide ukrainien de 1932 1933. La séance est suspendue.

La séance est reprise. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jean Derian qui fut sénateur des Côtes d'Armor, de 1997 à 1998. La parole est à madame Nadia Sollogoub pour une mise au point, au sujet d'un vote. Merci monsieur le président. Mon collègue le sénateur Bernard Delcros souhaiterait faire rectifier des positions de vote sur des scrutins publics concernant la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France sur les scrutins 280 cas, 285, 287 et 288, il a été noté comme compte en votant pour alors qu'il souhaitaient voter contre. Je vous remercie. Merci monsieur le président. Concernant le scrutin numéro 284 sur l'article 8 de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France mon collègue Julien Bargeton souhaiterait rectifier son vote pour voter contre et moi-même je souhaiterais rectifier mon vote pour vous m'abstenir. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Christian Vilac. Également pour une mise au point, sujet d'un vote. Merci monsieur le président. Dans ma mise au point concerne les scrutins. 284 285. 286, 287 et 288. Portable sur la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France. Mon collègue Stéphane Artano soit voter pour. Acte est donné de ces mises au point. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans la liste politique. Du scrutin concernés pas donc dont il y a une autre mise au point. Oui, sur le même sujet, donc on concernant le scrutin de 194 sur l'article 8, je vote également contre. Madame Cazebonne. Donc qu'on a pris acte de cette mise au point et elle sera aussi publié au Journal officiel. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restantes en discussion. De la proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérive des influenceurs sur les réseaux sociaux ont été publiés. Ces candidatures sont ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution relative à la reconnaissance du génocide ukrainien de 1932 1933 présenté en application de l'article 34 1 de la Constitution par Madame, Joëlle Gariod mais âme et plusieurs de ses collègues dans la discussion générale. La parole est à madame Joël Guerriau mesdames, auteur de la proposition de la injection pour 10 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues permettez-moi tout d'abord de saluer la présence annoncée dans ces prix de but de Monsieur Vadim Omelchenko ambassadeur d'Ukraine en France et de son conseiller politique. Olexander Schwyz. Au de là. Merci de vos applaudissements pour eux. Au-delà de cette présence qui nous sonore. Je voudrais surtout les remercier tous de leur engagement exceptionnel au service de leur pays et de ses relations avec le nôtre. Ils sont à l'image de leur peuple et à travers eux. Je voudrais saluer ce peuple ukrainien si vaillant qui nous donnent chaque jour des leçons de courage et de détermination dans la défense de leur valeur de nos valeurs de démocratie et de souveraineté et je tiens aussi à rendre hommage au travail de notre ambassadeur sur place, Étienne De Poncins de ses équipes et de tous les Français, élus, enseignants ou membres d'ONG humanitaires qui ont choisi de rester en Ukraine, malgré le danger, pour aider ce pays qui nous est si chère. Nous sommes donc réunis aujourd'hui, mes chers collègues, pour débattre, enfin d'une proposition de résolution sur l'Holodomor. Déposé au Sénat le 9 décembre dernier et co-signé par nombre de nos collègues et au 1er rang desquels Nadia Sollogoub président du club du groupe d'amitié France-Ukraine, que je salue, elle aussi pour son engagement sans faille en soutien à ce pays martyrisé. Il nous a fallu beaucoup de temps hélas pour arriver à la discussion par d'autres assemblées de cette proposition de résolution nous espérions que la France serait le premier pays à l'adopter, a adopté une résolution condamnant ce génocide perpétré contre le peuple ukrainien en 1932 33. Plusieurs autres résolutions déposées au Sénat après la nôtre ont été examinées avant l'Assemblée nationale a adopté elles-mêmes en mars une résolution sur l'eau de morts en tant que génocide, inscrite, deux mois après la nôtre mais même si je ne peux que regretter l'inscription tardive de notre proposition de résolution à l'ordre du jour de notre haute assemblée. L'essentiel est d'avancer et de voter cette résolution très attendue par nos amis ukrainiens. Elle avait je le rappelle était salué par le président du Parlement ukrainien notre estimé collègue Rouslan Stefantchouk qui nous avait fait l'honneur de s'adresser à nous. Le 1er février dernier. Depuis cette tribune de l'hémicycle et avait insisté sur l'importance pour les sénateurs français de la voter. Je me félicite donc que le Sénat puisse en débattre aujourd'hui et j'espère l'adopter après le Parlement européen, après l'Assemblée nationale le 28 mars et de très nombreux autres parlements européens notamment tchèque irlandais belges, allemands, polonais, Islande cela est essentiel car l'histoire nous éclaire toujours sur le présent et des parallèles évidents peuvent être faits entre la situation actuelle en Ukraine et celle d'il y a 90 ans. Rappelons que l'Holodomor extermination par la faim fait référence à la famine organisée par le pouvoir stalinien avec méthode et cynisme en 1932 33, en rétorsion aux tentatives de libération du peuple ukrainien réclamant dès 1917 la création d'un état démocratique indépendant face à la dictature du prolétariat voulue par la Russie bolchévique. C'est le peuple ukrainien, sa culture, sa langue et tout simplement son essence, que l'on a cherché à détruire chaque vie humaine perdue devait alors signé la victoire du totalitarisme. Soviétique sur un peuple trop épris de liberté et d'indépendance aux yeux du Kremlin, les millions de morts, certains historiens par le même de neuf millions. Hommes, femmes et enfants tout s'immoler au nom d'une idéologie mortifère, témoigne un par un, de l'horreur qui peut être déchaînée par un pouvoir sanguinaire pensante agir en toute impunité. Mal nommer les choses, c'est ajouter aux malheurs du monde disait Albert Camus. Alors oui, disons-le, il y a eu effectivement génocide car outre la famine systématiquement organisées dans les campagnes avec l'interdiction faite aux paysans de se réfugier dans les villes un peu mieux approvisionnés. Les exécutions systématiques des résistants et la déportation de centaines de milliers d'enfants en Russie pour les priver de leur identité et de leur langue, sont clairement constitutive de génocide. Raphaël M.. Le juriste international qui a défini les critères d'un génocide en amont du procès de Nuremberg dès 1948, avait qualifié cette Holodomor d'exemples classiques de génocide soviétique bien évidemment la Russie refuse de reconnaître cette qualification de génocide. Alors bien sûr cette reconnaissance d'un génocide ne mettra pas un terme aux malheurs frappant l'Ukraine du fait de son intolérable agression par la Russie de Poutine mais elle participera d'une part, atténuer les souffrances ukrainienne en leur manifestons notre indéfectible soutien, et d'autre part, à montrer à la Russie et au monde que nous ne sommes ni naïfs ni ignorants des faits historiques. Elle contribuera enfin à freiner la tentation russe de recommencer par ses actions inacceptables. C'est tout le sens des propos du président Zelensky qui commémorant les 90 ans de ce génocide dresser un glaçant parallèle entre hier et aujourd'hui, en déclarant le 26 novembre 2022. Autrefois, ils voulaient nous détruire par la faim aujourd'hui ils veulent nous détruire par l'obscurité et le froid incitant également les nations à faire état de leur soutien et de leur solidarité avec l'Ukraine en reconnaissant enfin l'Holodomor comme génocide. Nous ne saurions tolérer l'impunité et je me réjouis du soutien de la France réitérée par le président de la république dimanche soir à la mise en place d'un tribunal ad-hoc chargé de poursuivre les responsables des auteurs des auteurs des crimes d'agression contre l'Ukraine, comme l'Assemblée parlementaire de l'OTAN le réclamé dans une résolution dès mai 2022. Les auteurs de ces crimes ignobles que nous pouvons qualifier de terroriste devront répondre de leurs actes, tout comme comme nous, c'est, signons aujourd'hui devant l'histoire. Ceux qui ont perpétré l'Holodomor. Les chars collègue la dénonciation des atteintes aux droits humains des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a a toujours été au sein de cet hémicycle il ne ferme priorité qui nous rassemble bien au-delà des partis et des différences. C'est pour cela qu'à nouveau aujourd'hui. J'en appelle à votre sens de la responsabilité pour que nous soutenions de manière unanime cette résolution. Car reconnaître l'Holodomor comme un génocide, c'est s'opposer fermement aux forces du déni de l'indifférence et de l'injustice. C'est une déclaration de solidarité avec le peuple ukrainien qui lui offre la reconnaissance qu'il mérite pour soi résilience face aux tragédies si nombreuses et si actuelle ces tragédies qu'il a traversé tout au long de son histoire. Aujourd'hui. En Ukraine, si ce ne sont plus des drapeaux rouges qui flotte sur les ruines des villes martyres de l'Est ukrainien. Se sont bien à nouveau des décideurs terrés dans les alcôves du Kremlin qui organise l'agression de tout un peuple. Aujourd'hui les accablant témoignage qui nous sont relayées quotidiennement d'actes de torture, de viols et de cruauté commis par les troupes russes et les mercenaires sanguinaire de Wagner afin de briser la résistance du peuple d'Ukraine ne peuvent que que nous rappeler ces méthodes barbares employé il y a 90 ans par les autorités soviétiques. Aujourd'hui comme hier, à l'heure d'établir les responsabilités. Il nous faut faire résolument en face à la vérité et qualifié les faits aussi précisément que possible. Oui, je le répète, l'Holodomor est un génocide et présente toutes les caractéristiques détaillées à l'article 2 de la Convention pour la prévention des crimes de génocide de 48. À nouveau. Comme le 17 avril dernier, où vous savez chers collègues adopté à l'unanimité la proposition de résolution déposée par notre collègue André Gattolin qui condamné les transferts forcés d'enfants ukrainiens près de 740.000 selon les autorités russes ont Jules honneur d'être rapporteure je veux. Croire que la main du Sénat ne tremblera pas c'est pour cela que je vous exhorte aujourd'hui encore à voté solennellement et avec une même unanimité cette résolution à joindre vos voix, celles de nos collègues parlementaires de toute l'Union est de l'Ukraine, a rappelé avec force. Que nous n'accepterons jamais la tolérable et qu'hier comme aujourd'hui, ce qu'pensent pouvoir porter atteinte à l'humanité trouveront toujours sur leur chemin les représentants de la France, patrie des droits de l'homme nation des lumières et indéfectible soutien de la liberté des valeurs démocratiques partout dans le monde. Je conclurai en citant le texte d'une affiche ukrainienne de 1918, représentant une jeune paysanne ukrainienne protégeant son bébé et les champs derrière elle d'un vautour avec ces mots, je ne veux pas de ce qu'il ne m'appartient pas, mais je ne vous laisserai jamais me voler me voler ce qui est à moi. Alors, mes chers collègues, au nom de notre histoire et des valeurs qui sont les nôtres. Par respect pour le peuple ukrainien qui nous donnent chaque jour cet exemple de courage et de détermination et refuse de se laisser anéantir par plus gros et apparemment plus fort que lui, malgré les millions de morts de Lolo Rochefort et les tragiques perdent de beaucoup de ses enfants, aujourd'hui j'estime mes chers collègues, que nous avons un devoir moral de voter cette résolution pour l'Ukraine et pour nos valeurs et il en va de notre.

Aujourd'hui propose de reconnaître comme génocide l'Holodomor véritable extermination par la famine. Conduite par Staline et faisant plus de 4 millions de morts ukrainiens, soit 15% de la population entre l'été 1932 l'été 1933. Et ce. Alors même que la guerre fait rage en Ukraine. La méthode employée fut la terreur collectivisation forcée réquisition des récoltes. Russification à un fan. Déjà. Exécution. Autant de barbarie frappant la population ukrainienne à sans distinction depuis les paysages jusqu'aux intellectuels. Selon les historiens le régime stalinien. Ce dispositif dès 1929. Dans le but de véritables d'accaparer les richesses agricoles de Terrenoire ukrainienne en grande partie pour financer l'industrialisation rapide du pays tout en assurant le contrôle de cette république auto-soviétique. A donné à 600 toute velléité d'pas de l'Ukraine. Grenier à blé de l'Union soviétique. La famille ne fut la conséquence de l'extrême violence politique visant à briser les paysans Richard à la collectivisation à travers la. Je crois, sont des semences. Le blocus des villages. Par exemple pour ça la population jusqu'au cannibalisme, alors que là le même autant le régime continuaient d'exporter des tonnes de céréales ukrainiennes. Nul doute que ces crimes des journées constitue juridiquement. Génocide selon le droit international. Le président de l'Assemblée générale des Nations unies, rappelait récemment que le génocide est un processus graduel, les discours de haine. La déshumanisation des autres et l'évaluation récurrentes de leurs droits sont des précurseurs d'atrocités de masse. Le germe du génocide. Prolifère. Lorsque l'état de droit s'effondre. C'est un fait. Staline a organisé la termine de la pompe l'affaire ukrainienne entretenant méthodiquement la terreur, comme l'ont aussi fait d'autres. Génocidaires. Par exemple contre les Arméniens entre 1915 et 1923 contre les juifs lors de soit contre l'étude sur Rwanda en 94 ou encore au Cambodge ou Radek Yougoslavie. Aujourd'hui, 90 ans après les faits. 10 ans après le début du conflit dans le Donbass et l'annexion de la Crimée. Ça te pages sombres de l'histoire a ukrainienne résonne une actualité glaçante pour ce pays indépendant devenue le terrain d'une guerre totale depuis son invasion par l'armée russe le 24 février 2022. Or toute la guerre se joue aussi sur le terrain de l'information en l'occurrence. Celui de la désinformation. Le régime russe actuel n'a de cesse d'utiliser ce levier pour réviser l'histoire. Qualifiant les dirigeants ukrainiens de nazis. Les enjeux mémoriels autour de cette question n'assureront pas la victoire de l'État ukrainien aujourd'hui. Mais c'est aussi sur le terrain symbolique. Que les batailles semaine. Est-ce un hasard si le site de l'Assemblée nationale a été frappé par de cyber attaque. Revendiquée par des hackers russes le 27 mars dernier, veille des débats sur la reconnaissance de Holodomor comme génocide. Sans oublier. Ça le subir par le site internet du Sénat la semaine dernière. Je vois une motivation supplémentaire pour conduire les batailles sur le terrain mémorielle et exercer pleinement notre devoir de mémoire. Nous pourrons ainsi contribuer avec nos alliés à ce cours qu'une forme de révisionnisme ne Vienne effacer de l'histoire européenne. Ces crimes commis par le régime soviétique. Énième. Un marqueur démocratique fort pour toute cette en action et de reconnaître les crimes du passé afin de contribuer à faire qu'il ne se répète pas. Comme le rappelait mon collègue André Guyaux là sa tribune le 4 mai dernier. À propos de la résolution adoptée sur la réelle pour déportation par le pouvoir russe. De milliers d'enfants ukrainiens voter cette proposition de résolution. C'est répondre aux tentatives d'effacement de la mémoire collective. Car dans la guerre informationnelle qui se joue. Il est impératif de qualifier avec justesse les crimes commis hier. Comme ceux commis aujourd'hui. Alors. Suivant l'exemple du Parlement européen. Du Bundestag. De la Chambre belge et de nos collègues députés. Et votant cette résolution visant à qualifier de génocide. Les crimes barbares de l'Holodomor ukrainiens et à les inscrire dans l'histoire. Il en va aussi de notre devoir d'humanité. La parole est à monsieur Bruno Belin pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Sur le président chers collègues chez le ministre. Il est un abîme infernales. Une question diabolique que l'humanité aurait souhaité ne jamais se poser. Jusqu'où l'homme peut-il perdre. Certes, histoire de l'humanité a avant tout été sanglante et meurtrière. Mais si la chronique des millénaires relate avant tout une danse macabre d'escapades militaire le 20ème siècle fut le théâtre d'une sorte d'apothéose du mal avec ces massacres de masse. Ces crimes contre l'humanité, ces génocide. Cela a été dit, le martyre arménien la Shoah, la folie des Khmers rouges, le Rwanda, sans oublier l'Holodomor. Évidemment avant 1900 la cruauté et l'inhumanité ont pu aussi régner aucune terre n'a été épargné. Certainement pas notre sol de France. Ou la Saint-Barthélemy vit la scène devenir un fleuve de sang ou la terreur révolutionnaire et les colonnes infernales de Turow plongeurs la Vendée dans un bain de feu. Mais la spécificité maléfique des génocides du XXe siècle c'est leur organisation, leur planification l'horlogerie du Crime jusque dans la mise en scène de sa négation. Si nous sommes aujourd'hui réunis autour de cette résolution. C'est pour lever un voile et même un marbre obscènes qui recouvre cette page terrifiante du passé de l'Ukraine. Alors que certains hier d'autres aujourd'hui, refuse de reconnaître la réalité et l'intentionnalité de ces atrocités. Il est de notre devoir de rétablir cette vérité glaçante. En 1932 1933, des millions d'Ukrainiens avant tout paysans ont été condamnés à la mort par la fin. Si l'oubli est une seconde mort. Le déni est un second Crime. Oui, Staline et ses six cambre savait que la famille n'avait passé son noeud coulant sur les campagnes d'Ukraine. Oui, Staline et ces diables voulait éradiquer voir disparaître ces paysans et ils ont pris certaines décisions dans ce but. Le Petit Père des peuples a eu beau nier parler de fable pour rejeter les accusations ciseler une contre-propagande grossière avec des tournées mascarade. 2 personnalités occidentales comme Édouard Herriot, découvrant une Ukraine où tout allait bien. La guillotine sèche s'est abattue sur des millions d'Ukrainiens. On ne saura d'ailleurs jamais leur nombre exact. La guillotine sèche ses larmes du bourreau qui ne veut pas voir ses mains souillées du sang de ses victimes du bourreau ignoble et Tartuffe qui ose croire que son péché sera invisible, pas de sang, pas de crime. Si à l'instar de la Shoah. L'Holodomor n'a pas sa conférence de Wannsee. Il repose sur quelques décisions politiques sans aucune ambiguïté du gouvernement de l'URSS. La tristement célèbre loi des épis du 7 août 1932, qui punit de déportation ou de mort tout Vol ou dilapidation de la propriété socialiste ne serait-ce que par la simple appropriation de quelques épis dans un Champ 125.000 affamé malheureux seront condamnés dont 5400 à la peine capitale. Mais aussi les circulaires du 27 décembre 32 et du 22 janvier 1933, signant de fait les paysans ukrainiens à résidence et l'empêchant donc de fuir la famine. Et pendant ce temps cyniquement l'URSS de Staline exporter des millions de tonnes de céréales notamment ukrainienne pour financer son industrialisation à marche forcée. Les négationnistes, parmi lesquels de prétendus historiens très souvent idéologiquement marquée argue d'une famine bien réel qui frappait alors nombre de territoires soviétiques n'épargnant presque que les dignitaires du Kremlin et les responsables communistes ayant évité les premières purges. Mais une famine même largement répondu répandue ne serait ni excuser ni masquer la volonté. Délibérée d'extermination de découle accusations ukrainiennes. Personne ne doit désormais ignorer le témoignage. Contemporain du journaliste gallois Gareth Jones ressuscité en 2019 par le film bouleversant l'ombre de Staline Agnès cas Hollande ni les photographies de l'ingénieur Alexander une heure Berger. Mes chers collègues, l'Holodomor comme la Shoah et tous les autres génocides apparaît comme le mal absolu. Le refus même de la civilisation. Souvenons-nous du 5ème commandement du Décalogue tu ne tueras point met aussi du 8ème. Tu ne t'. Témoignera pas faussement contre ton prochain. Quand la nuit c'est de revenir, il faut allumer les flambeaux a écrit Victor Hugo à nous aujourd'hui dans cet hémicycle, comme d'autres parlementaires européens pu le faire de servir non pas le devoir mais l'impératif de mémoire et de vérité. Je vous remercie. Dans la suite de la discussion, la parole est au président Claude Malhuret, pour les indépendants pour cinq minutes. Nous ne savions pas. Combien de fois cette excuse a-t-elle servi à ceux qui ont choisi de fermer les yeux. La Shoah, elle avait lieu dans le secret des quand. Le génocide khmer rouge dans un pays cadenassé l'Holodomor dans l'Ukraine impénétrable. Le goulag dans l'inaccessible Colima le là-haut Gail au fin fond de la Chine interdite. Cette excuse je n'y crois pas. La vérité ne s'est jamais dérobé qu'à ceux qui ne voulaient pas voir. Ces massacres ces génocides ces crimes contre l'humanité ont leur bourreau. Mais aussi leurs complices. Les bourreaux sont connus de Hitler à Staline de Mao à Mengistu de Pol Pot aux généraux birmans. Là où nous sommes concernés. Ce sont les complices. Les complices actifs d'une part les idiots utiles de l'autre. Les complices chez nous en 39 45 les fascistes français et les collabos. Du temps de l'URSS, les partis communistes occidentaux flanqué le temps d'intellectuels prestigieux du temps des 40 millions de morts du grand bond en avant les sectes maoïste puissamment aidé par la fine fleur de l'intelligentsia française. Les idiots utiles. Écoutez-les pendant l'Holodomor Édouard Herriot qui en revient. Elle était 33, je vous affirme que j'ai vu l'Ukraine-t-elle un jardin en plein rendement, il n'y a que jardin potager et. Admirablement irriguer cultivé et récolte décidément admirable. Des phrases aussi inimaginable ont été préférés proférées par des Romain Rolland des Langevin des Malraux et des dizaines d'autres. Toutes ces visites Potemkine ont eu lieu au plus fort de la famine lorsque des parents mangé leurs enfants morts lorsque la loi sur les épis, condamné à 10 ans de camp ou à la peine capitale. Toute personne ayant glané quelques épis de blé ou de seigle dans les champs. De toutes les victimes des génocides, des famines organisées des massacres, certaines ont été victimes de fois une première fois. Une deuxième fois lorsque les crimes n'ont pas été jugés les bourreaux qui ont perdu ont été condamnés parfois avec beaucoup de retard mais condamné les nazis à Nuremberg. Les Khmers rouges à Phnom-Penh les génocidaires hutus à La Haye. Mais il n'y a pas eu de Nuremberg. Pour ceux qui n'ont pas perdu leur guerre les Staline les Mao Tsé-Toung et tant d'autres sont morts dans leur lit. Pire, ils ont eu tout le temps de maquiller l'histoire et de s'exonérer. Seuls les historiens peuvent les juger et c'est si difficile lorsque les preuves ont été effacés. Combien d'années a-t-il fallu pour tribut à Staline l'Holodomor le massacre de Katyn le goulag pour enfin connaître le bilan du grand bond en avant en Chine. Pourquoi faut-il que ces forfaits soient condamnés même longtemps après pour la mémoire des victimes bien sûr mais pas seulement. Pour tenter d'éviter aussi de nouvelles atrocités, je dis bien tenté. Car malheureusement, l'histoire se répète. 90 ans après l'Holodomor l'Ukraine perd des centaines de milliers de ses enfants par le Crime d'un ancien colonel du KGB devenu le dictateur fasciste du Kremlin et les mêmes complices et les mêmes idiots utiles sont là si je parle de. C'est parce que je les connais. Je les ai rencontrés tout au long de ma vie en 1980 lorsque Médecins sans frontières a organisé la marche pour la survie du Cambodge pour dénoncer la famine organisée par les Vietnamiens. Nous avons fait face à une campagne internationale expliquant que nous étions des agents de la CIA en 1984 lorsque nous avons dénoncé les déportations de masse en Éthiopie. Nous avons été traités de menteurs, non seulement par Mengistu mais par l'attelage improbable de plusieurs ONG de l'ONU et même du misérable, ambassadeur de France, des années plus tard, une fois renversé Mengistu sera condamné pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et abrité au Zimbabwe par son ami le dictateur Mugabe il coule aujourd'hui des jours paisibles à Harare. D'autres exemples ne date pas d'hier mais d'aujourd'hui. Les Ouïgours les Rohingyas les massacrer de l'Est du Congo, ceux de la République centrafricaine avec l'aide des ordures du groupe Wagner dans l'indifférence générale et le négationnisme des complices et des idiots utiles. Aujourd'hui, l'Ukraine est victime de nouveaux crimes contre l'humanité, presque aucune des résolutions prises à l'Assemblée, au Sénat ou au parlement européen condamnant la guerre de Poutine n'a été voté ni par le Rassemblement national ni par les insoumis ni par le parti communiste le 28 mars dernier, l'Assemblée nationale a voté contre comme nous aujourd'hui une résolution sur l'Holodomor. La France insoumise a refusé de participer au vote, le parti communiste a voté contre. C'est un nouvel affront infligé à la mémoire des millions de victimes de Staline mais aussi de celle de Poutine. Merci à notre collègue Joël Guerriau mais la face aux falsificateurs de l'histoire, le Sénat sonore aujourd'hui de célébrer la mémoire des victimes de l'un des pires crimes du XXe siècle. Demain, après la victoire de l'Ukraine. Il faudra que se tienne le Nuremberg du poutinisme et de ses complices. Merci cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est à monsieur au président Guillaume Gontard, pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour cinq minutes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre. Le 26 novembre dernier, les Ukrainiens et ukrainiennes commémorer le 90ème anniversaire de la grande famine. La grande famine a entraîné la mort de plusieurs millions de personnes entre 1932 et 1933 en République ceci socialiste soviétique d'Ukraine. C'est en 1920 que le dirigeant de l'URSS Joseph Staline décide de lancer la collectivisation forcée dans le but d'ouvrir des fermes d'État. Les Terres et les productions des paysans sont confisqués les prélèvements sur les récoltes continue à augmenter de manière disproportionnée. Alors que des familles éclate dans plusieurs pays, comme au Kazakhstan. En réaction à la politique meurtrière de Staline, des actes de protestation et de contournement des règles s'organisent partout. L'Ukraine et en particulier ces paysans compose au coeur de cette résistance. Pour briser cette résistance Staline et son gouvernement décide de durcir encore leurs mesures pour aggraver la famine. Les villages affamés sont isolés et les paysans n'ont pas le droit de gagner les villes entre 3 5 et 5 millions de personnes mourront dans des conditions atroces. Cet épisode de la politique meurtrière de Staline porte le nom de l'eau de mort qui signifie littéralement extermination par la faim en ukrainien. car pour beaucoup pardon d'l'historien l'intention de Staline était bien avec cette politique criminelle d'anéantir les Ukrainiens. Aujourd'hui la Rada ukrainienne nous demande de reconnaître la grande famine comme un génocide du peuple ukrainien. Car la grande famille est un épisode de l'histoire qui fait aujourd'hui partie intégrante de l'identité ukrainienne. Pendant plusieurs décennies. Les autorités soviétiques ont tenté d'étouffer la vérité. En vain car la vérité n'est pas une opinion. C'est en 2004 après l'élection de Viktor Iouchtchenko, que le peuple ukrainien. Dénonce les actes barbares et meurtrier de Staline en 2006, 74 ans après la grande famine. L'Ukraine élève l'Holodomor au rang de tragédie nationale puis reconnaît comme génocide. Depuis. De plus en plus d'États reconnaissent la grande famine comme génocide l'Allemagne l'a fait au mois de novembre dernier et le parlement européen au mois de décembre dernier. Les Ukrainiens et les Ukrainiennes n'ont pas eu la possibilité en 2022 de commémorer comme il se doit ce 90ème anniversaire. Pas de grands rassemblements seulement des cierges allumées aux fenêtre et une minute de silence. Car, comme nous le savons tous. Depuis le mois de février 2022, le peuple ukrainien est de nouveau attaqué. Si le régime a changé. L'agresseur est le même, le voisin russe qui a toujours la plus grande difficulté après des siècles d'histoire partagée à accepter l'existence même de la nation ukrainienne. Les intentions de Vladimir Poutine quand il a envahi son voisin. Il y a 15 mois ne faisait aucun doute. Annexion de l'Ukraine ou a minima, mise en place d'un pouvoir fantoche, la colonne de chars envoyés sur Kiev en février 2022 illustrent cette velléités impérialistes. Ils bombardent des civils torture il attaque des établissements médicaux. Et nous en avons débattu récemment dans cet hémicycle il enlève des enfants. La logique de ces atrocités et toujours la même, faire disparaître la nation l'identité nationale ukrainienne, ses enfants, dont le nombre est estimé à 16.000 sont déportés en Russie puis emmenés dans des camps de rééducation qui ont pour but de les endoctriner en les noyant dans la propagande pro-russe et dans les entraînements militaires Poutine cherche ensuite à faire adopter ses enfants ukrainiens par des familles russes. Le massacre de Bubka villes ukrainiennes, dont l'armée russe s'est retiré il y a un an, porte encore les stigmates de cette volonté d'anéantir la population ukrainienne. Lors du retrait des troupes russes. Les soldats ukrainiens ont notamment découvert dans cette ville, des dizaines de corps de civils vraisemblablement exécutés. Mais Vladimir Poutine comme Joseph Staline avant lui commet une erreur fondamentale. Considérer que l'Ukraine n'est qu'un territoire riche en ressources, notamment céréalière, dont la Russie peut disposer à sa guise sont les besoins de son pouvoir central. Cette idéologie de faussaires de l'histoire, ignore la construction nationale ukrainienne, qui s'est affirmée depuis 2 siècles avec autant de force que toutes les autres nations européennes. en menaçant pardon jusqu'à son existence. Vladimir Poutine ne fait que renforcer l'identité nationale ukrainienne et plus qu'à d'autres périodes de son histoire, la pousse vers l'ouest du continent. Il est de notre devoir d'Européens d'accompagner ce droit du peuple ukrainien à disposer de son destin. La reconnaissance du génocide ukrainien en fait partie. Elle n'est pas aussi efficace que notre soutien militaire, financier et humanitaire, elle revêt une importance symbolique dont il ne faut en aucun cas négligé la puissance en votant cette révolution cette résolution pardon nous exprimons une nouvelle fois notre solidarité sans faille à l'Ukraine et à son peuple. Merci. Dans la suite de la discussion, la parole est à madame Nadège avait pour le groupe RDPI pour six minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Reconnaissance envers les députés de l'Assemblée nationale pour cette décision historique. C'est par ces mots postés par le sur les réseaux sociaux que le président Zelensky avait réagi au vote du 28 mars dernier en faveur de la reconnaissance et de la condamnation de l'Holodomor comme génocide. Cette proposition de résolution déposée par la députée Anne Genetet et nombre de ses collègues porter de façon transpartisane est adopté à la quasi-unanimité invité le gouvernement français à reconnaître officiellement et a condamné publiquement le caractère génocidaire de ces crimes de masse commis à l'encontre du mot peuple ukrainien. Il y a 90 ans. À la signature à l'initiative, pardon de la sénatrice Gariod Mélane dont je salue la proposition, notre haute assemblée s'apprête à son tour a formulé une demande identique. Reconnaître et condamner officiellement la famine la déportation et l'extermination méthodiquement organisé par les autorités soviétiques à l'encontre de millions d'Ukrainiens en 1932 et 33 Le groupe RDPI votera ce texte qui fait suite à 2 autres votes intervenus depuis le début de l'année là en faveur de la résolution de notre collègue Claude Malhuret en février dernier où nous avions alors exprimé le soutien du Sénat l'Ukraine condamner la guerre d'agression menée par la Fédération de Russie depuis maintenant plus d'un an et a appelé au renforcement de notre aide, l'autre en soutien à la résolution européenne du 17 avril déposée par André Gattolin où nous avions condamné les déportations d'enfants ukrainiens par la Fédération de Russie. Les souffrances d'hier font écho à celles d'aujourd'hui. Alors que les années 2022 2023 consacrent, je le disais, le 90ème anniversaire de l'une des plus grandes tragédies du siècle dernier. Le texte qui nous est soumis, cet après-midi répond à un appel fait au Parlement des nations qui soutiennent l'Ukraine. Celle-ci a été formulée en octobre dernier par le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Dmytro Kuleba qui repris par le Parlement ukrainien pour de la reconnaissance du caractère génocidaire de Lolo de morts. Ce texte ce terme ukrainien qui se traduit par extermination par la faim désigne la grande famille qui a sévi en début des années 1930, entraînant la mort de plusieurs millions d'Ukrainiens cette famille politique et non climatique d'une ampleur effroyable a été orchestrée par Staline entre 1930 et 1933 sur plusieurs régions de l'URSS, parmi lesquels l'Ukraine dès la fin 1929 a été initié la. Collectivisation forcée des Terres et s'est accompagnée d'une campagne de répression en Union soviétique dirigée contre les coups La Hague les propriétaires terriens. Avec des expropriations des arrestations de déportation et d'exécutions massives en lieu et place ont été instaurés des entreprises agricoles. Collective des sauf. Des kolkhozes placée sous l'autorité de l'État, un système de réquisition a alors été mise en place, provoquant le soulèvement et la révolte de la paysannerie ukrainienne. La réponse répressive des autorités soviétiques a été immédiate et des brigades ont été dépêchés contre les émeutiers, les récoltes ont été confisqués. Les conséquences sur 10 désastreuse, provoquant un exode rurale de masse en réaction d'entrer dans les villes fut empêché un blockhaus instauré avec encore des arrestations et des déportations en Sibérie et dans les camps du goulag, avec de nouveaux des mesures confiscatoire, à savoir le retrait des produits manufacturés et alimentaire et des impositions exceptionnelle. La loi des épis fut programmé le 7 août 1932, perdant mettant de condamné à 10 ans de camp ou à la peine de mort tout Vol ou dilapidation de la propriété socialiste. Des milliers de paysans ukrainiens mourraient chaque jour affamés alors que même dans le même temps, plusieurs millions de tonnes de céréales ukrainiennes étaient alors exporter. Après la chute de l'URSS et l'ouverture à de l'accès à certaines archives le voile sur cette période dramatique, a été levée une atrocité pourtant à nouveau réfuté par Vladimir Poutine en 2006 sur la base d'un consensus au sein de la population concernant cette qualification de ce Crime de masse le Parlement de l'Ukraine, a reconnu la famine comme génocide contre contre le peuple ukrainien dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Le 15 décembre dernier, le Parlement européen également à travers une résolution est venu reconnaître le caractère génocidaire de l'Holodomor. Nous soutenons avec mon groupe, la demande qui est faite à la France de suivre cette voie par cette proposition de résolution, il s'agit pour nous de proclamer l'indéfectible attachement de la France au respect de la dignité humaine d'exprimer une nouvelle fois le soutien du pays au peuple ukrainien en reconnaissant les atrocités les souffrances qu'il a subi dans son histoire par cette proposition de résolution, il s'agit de condamner cette volonté répétée de négation de l'identité et de la nation ukrainienne. Je veux reprendre les propos tenus en explications de vote à l'Assemblée nationale fin mars. Voter pour cette résolution c'est aussi confirmé aux Français aux Européens et au monde que lorsque les Wagner essentielles et universelles sont en jeu, il n'y a ni majorité ni minorité ni centre ni droite ni gauche. Mais oui un Parlement qui représente la nation toute entière et qui votent en conscience, je vous remercie. Merci cher collègue. Dans la suite de la discussion, la parole est au président Kanner pour le groupe socialiste, écologiste républicains pour cinq minutes. Applaudissements Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, La famine qui a été organisée par le régime stalinien entre l'hiver 32 et 33 est une abomination. Qui a fait plusieurs millions de morts, les chiffres ne sont pas vraiment arrêter. Cette année ayant pris soin d'interdire la divulgation des chiffres du recensement de 37 trop par l'armistice. Divulgation donc n'était pas possible. Mais pourtant, nous pensons qu'. Il y avait entre 5 et 7 millions de paysans qui ont disparu dans les conditions qui ont été rappelés déjà à plusieurs reprises. Ukrainiens de souche pour la plupart. Qui ont péri dans ce terrible épisode le grenier à blé de l'Union soviétique était devenue sa fosse commune. Le pouvoir soviétique avait réquisitionné toutes les récoltes de la région et jusqu'aux moyens de production, de la nourriture afin de créer une famine artificielle d'où le nom de l'eau de morts. Des déportations des tortures physiques ont également été commises lors de cette période mais je ne reviendrai pas sur l'ensemble de ces faits ma collègue Hélène commémorer qui va bientôt s'exprimerait s'exprimer il reviendra. Ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui c'est la volonté de Staline derrière cette décision en ciblant plus particulièrement les paysans ukrainiens étaient affirmé la volonté d'éradication de l'identité ukrainienne et du Patrimoine qu'pouvait comporter afin de contenir toute velléité de contestation du joug soviétique. La guerre des mémoires qui fait rage sur la scène internationale depuis plusieurs décennies entre l'Ukraine et la Russie nous montre les enjeux identitaires qui se cache derrière ce ce ce génocide pardon. Certes, l'histoire ne se répète pas mais elle éclaire le présent. Sans revenir sur l'ensemble de ces enjeux. Il est aisé de comprendre que l'Ukraine s'est émancipé de la sphère culturelle des slaves de l'Est dans laquelle Moscou souhaiter la circonscrire. Et qui était en victime de l'oppression soviétique le peuple ukrainien s'affirmer nécessairement comme intrinsèquement autre. La Russie quant à elle reste assise sur une identité empreintes des prouesses passées et notamment l'industrialisation à marche forcée des années 30 qui permit notamment la victoire contre l'Allemagne nazie. Personne ne peut le contester. Le terme de génocide, établissant un parallèle entre Staline et Hitler. L'on comprend que Moscou ne pouvait l'accepter sans remettre en cause les fondements de sa propre identité l'de morts, devait être dénoncé comme l'un des crimes les plus stalinien. Des crimes les plus horribles de l'histoire stalinienne. C'est ce que nous faisons aujourd'hui ne pas le reconnaître ce réécrire ou déformé l'histoire. Les parallèles qui peuvent être faits avec la situation actuelle sur notre continent et dans notre pays sont nombreux. La résonance avec la guerre qui sévit actuellement en Ukraine est nécessairement saisissante. Par ailleurs, l'Holodomor ne s'est produit qu'à quelques centaines de kilomètres de la frontière cette proximité doit être également. Revisiter ma première source d'inquiétude que je tenais à exprimer devant vous aujourd'hui, vient de la mort de la montée du nationalisme en France. Qui conduit systématiquement à des violences. À une vision hégémonique voire suprémacistes d'une identité par rapport aux autres. Les dangers du nationalisme en France n'ont jamais été aussi prégnant qu'actuellement. Le déferlement de la violence de l'extrême droite en particulier. On est une preuve, on l'a évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure dans le cadre des questions d'actualité au gouvernement. Il y a une totale désinhibition que ressent aujourd'hui l'extrême droite dans notre pays et qui exprime sans contrainte c'est plus sombres position. Nous devons donc être vigilants à ce que les nationalismes ne gagne pas ou plutôt devrais-je dire ne gagne plus notre continent. Le de morts. Doit être reconnu comme l'un des 3 crimes contre l'humanité les plus marquants du XXe siècle avec le génocide arménien et l'holocauste et, plus loin de nous peut être le Rwanda même sûrement le Cambodge et d'autres exemples qui ont été cités par nos collègues. La proposition de résolution. J'remercie son auteur qui nous est soumis, qui est soumis à notre examen fait appel à notre devoir de mémoire. Elle est à saluer. Je pense que ce devoir de mémoire doit aujourd'hui passer un devoir de vigilance au regard des enseignements du passé. une vigilance accrue car les heures sombres ne sont jamais très loin alors que le nationalisme exacerbé et le populisme s'entremêlent. Le groupe socialiste, écologiste et républicain votera cette proposition de résolution de nos collègues et se rappelle un douloureux passé. Doit nous inciter. Monsieur le Ministre à ouvrir dès que possible les portes de l'Europe au peuple ukrainien. Je vous remercie. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à la fin des années 20. Staline rompt avec la nouvelle politique économique établi en 1921 dans la nouvelle union soviétique. Il décide alors d'engager une collectivisation forcée des Terres agricoles à un rythme effréné et avec une brutalité inouïe. Cette décision va désorganiser durablement et en profondeur les récoltes et la paix sera Nery au seul profit de la constitution d'une industrie lourde. Le coût humain on fut terribles dans toute l'Union soviétique, en particulier dans les années 1932 1933. Ou après de terribles récoltant 31 et 32, les quotas imposés prélevées par l'État ne furent corriger qu'à la marge. Oh Gendron des familles historiques. Dans sa quête fanatique de ses objectifs économiques le pouvoir stalinien et ses relais locaux iront jusqu'à établir des blocus afin que les agriculteurs ne déserte pas les Terres. Tout particulièrement en Ukraine. Ce sont des millions de citoyens soviétiques ukrainiens mais aussi kazakh et russe, qui en furent victimes. L'Ukraine fut particulièrement frappée, selon l'historien craignant de référence Stanislas coucher ski ce sont 3 à 3 millions et demi de personnes en Ukraine qui décède suite à cette famine dans une étude de démographes ukrainien de 2008 le nombre de morts excédentaire en Ukraine pour la période de 1926 à 1939, c'était deux 3 millions et demi. Dont la plupart durant les famines du début des années 30, ces famine de l'ère soviétique produisirent davantage de victimes que la grande famine russe de 1891, 1892. Et plus encore que les familles n'résultant de la guerre mondiale et de la guerre civile. C'est d'ailleurs notamment pour conjurer ses famines que la NEP avait été établie en 1921. Avant l'ouverture des archives de l'URSS la théorie. Intonations intentionnalité selon laquelle Staline avait consciemment tué par la fin. Les paysans ukrainiens parce qu'ukrainien était répandue depuis le début des années 2000, le travail des chercheurs a réouvert le débat Roland Davies Stéphane Crop marteau guerre et Hiroki Kuriyama qui ont travaillé sur les archives et les correspondants des dirigeants de l'époque mettent en cause cette thèse. De qualification de génocide en 2022 lors de l'examen du débat sur une résolution traitant elle est elle aussi de l'Holodomor le Parlement belge, a sollicité l'avis d'historiens qui ont considéré ce terme inapproprié pour désigner ces familles l'historien français Nicolas Werth qui lui, admet le terme de génocide. Expose dans une tribune récente au monde l'objet et l'existence de ces débats d'historiens. La qualification de génocide continue donc de faire débat. Ce débat n'atténue pour nous en rien ni l'ampleur des crimes commis contre la paysannerie de l'époque ni la terrible responsabilité du pouvoir stalinien dans ce drame abominable. D'autant que s'y ajoutaient une cruelle répression envers ceux qui étaient considérés comme des opposants qui décima d'ailleurs est également massivement les rangs des communistes. La dit la dénonciation de ces crimes staliniens et pour nous irrémédiable. D'autant que face à l'ampleur de la famine effrayé de montrer la réalité Staline mis sous scellés les informations là révélant empêchant toute solidarité nationale ou internationale aggravant considérablement ses effets. Les sénateurs communistes tiennent par ailleurs à interroger l'intention politique de cette résolution nous avons voté la dénonciation du Crime de départ tation d'enfants ukrainiens. Il y a quelques jours, nous n'avons pas chez rapportrice la main qui tremble. J'imagine que les auteurs de cette résolution souhaite à travers son adoption apporter une marque de soutien à l'Ukraine. Et je l'espère à la perspective d'une paix civile retrouvée à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières ukrainiennes. Or il est Or il est frappant de constater que la guerre des récits nationaux et depuis 10 ans au coeur. Du conflit. Poutine ne cesse de réécrire l'histoire pour justifier sa croisade criminelle au nom d'une prétendue dénazification en Ukraine des responsables. Il serait. Réhabilite Stepan Banderas en effaçant les les épisodes plots glorieux de son histoire. Comme si la guerre d'aujourd'hui était était condamnés à répéter les crimes du passé. la chute de l'Union soviétique continue de réveiller des frontières, non seulement physique mais pouvez historique, culturelle, politique et mémorielle qui nourrissent les conflits d'aujourd'hui. Et que la construction d'une Ukraine en paix dans ses frontières étatiques. Devra dépasser pour faire vivre ensemble l'entièreté de sa population. Est-ce notre responsabilité d'alimenter au coeur de la guerre actuelle. Ces conflits mémoriels Hélène qu'ils alimentent. Cette résolution nous son nom que relever moins d'une reconnaissance historique et d'une compassion légitime à l'égard des victimes de la famine. Qu'au souci d'alimenter le récit de justification de l'amplification de l'effort de guerre réclamée par les dirigeants ukrainiens au détriment de la recherche d'une reconstruction de la paix. Pour toutes ces raisons et aussi pour exprimer plus généralement notre malaise face à l'inflation parfois inappropriée du Khalek qualificatif de génocide par définition. Et exceptionnelle dans le cadre de résolutions parlementaires. Le groupe CRCE votera contre cette résolution. Merci cher collègue. Dans la suite de la discussion. La parole est à monsieur François Bonneau. Pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La famille orchestrée par l'URSS. Entre 1932 et 1933. Nous rappelle la difficile construction l'identité ukrainienne longtemps oppressé aujourd'hui menacés par la Russie. La population ukrainienne répartis dans la région de l'Ukraine actuelle et du coup bon a été forcé de collectivisé les Terres agricoles afin de permettre l'industrialisation de l'empire soviétique. Le plan de collecte élaboré par Staline a engendré des ponctions de plus en plus importante des récoltes au détriment de la population ces dernières étaient de l'or, de 30 pour 119.130, pour atteindre plus de 55% à partir 1932. Face à l'opposition virulente des responsables communistes ukrainiens et de la population le régime soviétique à utiliser l'arme de la faim pour briser le mouvement paysan. Ce châtiment par la enfin visait en réalité à éteindre l'identité nationale ukrainienne. Qui revendiquait déjà. Son indépendance au moment de la révolution bolchévique. Leur droit à disposer d'eux-mêmes avaient été proclamée par la Rada central et une première insurrection paysanne à brouiller les plans de conquête bolchévique de l'Ukraine. Au printemps 19. Des preuves d'intentionnalité du génocide ont été découvertes lors de la chute de l'empire soviétique. Les réserves de nourriture des paysans ont été confisqués et ils ont été condamnés à mort ou déportés. Le régime stalinien également empêcher l'exode des Ukrainiens qui ont tenté de fuir. Et mis un terme aux politiques d'Ukraine Isaksson. Ces preuves tangibles montre qu'il ne ça si ne sais, pas uniquement d'un Crime de masse mais bien d'un génocide, au sens de la Convention des Nations unies de 1948. Ce grenier à blé disposant des Terres les plus fertiles au monde, est devenue un charnier où une famille orchestrée fit disparaître dans d'atroces conditions, hommes, femmes enfants dont ne pouvons taire le Crime. de morts, ça a été dit que signifier tué par privation en ukrainien a fait entre 3 et 6 millions de victimes. Cet événement est d'un des socles de la reconstruction étatique national et identitaire de l'Ukraine post-soviétique. En 1986, Robert Conquest, un historien britannique a publié sanglante moisson qui explicite la machine génocidaire stalinienne. Son objectif était d'éveiller la conscience publique face à ce drame occulté et ainsi l'ancrée dans la mémoire collective. En novembre 2006, le Parlement ukrainien a reconnu la famine comme année génocide perpétré par l'URSS. À ce jour, 31 pays reconnaissent Holodomor comme un génocide. Le 15 décembre dernier, le Parlement européen a adopté à la quasi-unanimité, une résolution en ce sens, tout comme l'Assemblée nationale le 28 mars 2023. Nous ne pouvons pas rester insensible à cette tragédie. L'histoire nous montre une nouvelle fois combien ignorer et méconnaître ces faits n'est pas possible pour une nation comme la nôtre qui défend les droits humains, la paix et la liberté. La reconnaissance de ce génocide par la France est nécessaire afin de de mettre en lumière une politique d'assimilation et de destructions menées sur des populations civiles. L'invasion russe est venu raviver cette période dramatique pour l'Ukraine et sa volonté de maîtriser son destin malgré toutes les souffrances endurées. L'humanité ne peut pas vivre éternellement avec dans sa cave. Le cadavre d'un peuple assassiné comme le disait Jean Jaurès sur Metz. Merci cher collègue. Dans la suite de la discussion. La parole est à monsieur Jean Louis Masson pour le le groupe des non inscrits pour 3 minutes.

Je ne voterai pas cette proposition pour 2 raisons. Tout d'abord les faits ne correspondent pas à la définition juridique d'un est un génocide. Ensuite ma seconde raison est que cette proposition source a surtout pour but de nuire à la Russie. Or, tout s'est passé à l'époque de l'URSS et les vrais responsables sont les dirigeants communistes. Aussi bien ukrainiens que russes ou autres, n'oublions pas que Staline était géorgien que Khrouchtchev été ukrainien d'ailleurs au prorata de la population Staline a fait plus de morts au Kazakhstan qu'en Ukraine. Il faut donc une certaine mauvaise foi pour vouloir reporter les accusations sur la Russie d'aujourd'hui. C'est comme à Lucie à l'issue de la première guerre mondiale, lorsque les vainqueurs au prétendu que le seul responsable. On était l'empereur Guillaume II. C'est totalement faux car la cause de cette guerre fut l'assassinat de l'archiduc d'Autriche par des terroristes Serbes et. Les pays qui les soutenait à l'époque ont donc une large part de responsabilité, de même aujourd'hui les vrais responsables de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ce ne sont pas ces 2 pays ce sont au moins pour partie le trio des provocateurs l'OTAN les États-Unis et l'Union européenne. Lorsque l'URSS s'est effondrée. La disparition du Pacte de Varsovie aurait dû avoir pour corollaire la dissolution de l'OTAN. Hélas, en totale violation des engagements pris. L'Union européenne et l'OTAN se sont étendues vers l'Est y compris sur des territoires qui avait appartenu pendant, pendant des siècles à la Russie historique. À juste titre. La Russie s'est donc senti encerclé. Par le passé. Les États-Unis étaient prêts à engager une guerre nucléaire lorsque l'URSS a seulement voulu installer des fusées à Cuba. Aujourd'hui, c'est que le trio des provocateurs fait en encerclant la Russie et 10 fois pire que l'installation d'éventuels hypothétiques fusées à Cuba. C'est pour cela que je suis tout à fait hostile à l'adhésion de pays de l'ancienne URSS à l'OTAN et à l'Union européenne, laquelle n'est rien d'autre que le cheval de Troie de l'OTAN. Si la guerre reste conventionnelle. La Russie nie finira par s'effondrer farce face aux énormes moyens mis en oeuvre par les pays de l'OTAN. Le président Poutine acceptera-t-il alors que son pays soit humilié et militairement asservis. Par l'hégémonie de l'OTAN. Son seul choix serait entre se laisser écraser ou engager une escalade nucléaire. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir utilisé la bombe atomique alors même qu'ils étaient en train de gagner la guerre contre le Japon. Si la Russie est en train de perdre la guerre et si son existence est en jeu. Il se pourrait qu'elle décide d'utiliser tous les moyens dont elle dispose pour se défendre. Les États-Unis seraient alors mal placé pour lui donner des leçons. Merci cher collègue. La parole est à monsieur Bruno Belin pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. D'abord je tiens à saluer. Notre collègue Joël Guerriau. Auteur de cette résolution. Je voudrais aussi adressé un message. Fort de gratitude par rapport à l'action que mène la présidente du groupe d'amitié France-Ukraine ça honore ce Sénat merci à à Nadia et je voudrais évidemment salué l'ambassadeur, présent dans les tribunes et lui dire notre solidarité face à la situation du pays qu'il représente. Mais quand nous avons un tel texte ça a débattent, mes chers collègues, ce n'est pas sûr de l'affectif. Que nous devons évidemment nous. Basée et bien évidemment sur les faits et sur le droit international. Le droit international c'est la résolution de l'ONU de 1948 qui définit un génocide. On a évidemment en tête. Le génocide arménien la Shoah, le Rwanda au milieu des années 90, mais effectivement. Le droit international. Donne le cadre. Il y a l'intention. La volonté de détruire. Et la notion de groupe national, qu'ils soient religieux, ethnique ou raciale. Et si ces conditions qu'il faut évidemment regardée. Quand on passe de l'histoire et les faits. Bien sûr il y avait intention de détruire. Bien sûr il y avait intention nous sommes face à une barbarie organisée l'histoire raconte les faits. Il y a cette volonté de du leader soviétique dans les années 20. Il y a ce grand tournant puisque cette expression date de 1930 pour arriver à la situation connue de 1931 1932. L'arme de la faim contre les paysans ukrainiens. C'est ça le donnant et c'est est vrai que C'est dommage que la présidente assassine soit pas rester, je lui aurais mis au défi de regarder 2 fois de suite le film sur le nombre de Staline. J'ai essayé, c'est pas possible il y a un moment donné. Les faits sont là, évidemment. Ils sont poignants. Les les notions de cannibalisme ont été rappelés mais. C'était un tel point que même le régime soviétique, qui avait fait une affiche pour dire. Manger son enfant est un acte barbare. Alors il y avait bien effectivement cette notion de détruire. Mais il y avait bien cette volonté effectivement. D'anéantir la résistance des paysans ukrainiens. De grenier à à grains. L'Ukraine était devenue terre de sang et c'est là où on est finalement dans la 3ème notion du droit international le groupe national. Oui il y avait volonté de d'exterminer une partie du territoire soviétique. Alors bien sûr dans le débat, j'ai bien entendu les propos de certains de nos collègues. Il n'y avait pas que les Ukrainiens. Mais il y a eu à hauteur de 6, 7 millions cette volonté d'anéantir le peuple ukrainien. 31 pays ont d'ores et déjà. Reconnu ce génocide et je crois que nier c'est tuer une 2ème fois et ça sera l'honneur du Sénat français d'adopter cette résolution reconnaissant le génocide ukrainien. Je vous remercie. Dans la suite de la discussion. La parole est à madame Hélène comme ouais commémorer pour le groupe socialiste, écologiste républicains pour 4 minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La mémoire d'une douleur et toujours personnelles intime et le débat qui s'ouvre cet après-midi n'y échappent pas. Pour avoir vécu 30 en Irlande. J'ai le souvenir sur la côte ouest de l'île de cette vallée roux c'est vide où le regard ne s'accroche qu'à la seule croix de granit dédié à la tragédie de, d'où

Il est vrai qu'un jour de mars 1849. Plus de 400 personnes sont mortes de faim dans ce comté de Mayo lors d'une dernière marche qui leur avait été imposé par une une administration coloniale distribuant un secours d'urgence trop rare à des populations abandonnées. Elle vous taire ce faisant au million et demi de morts que qui la grande famine. Mon souci n'est pas cher collègue de relativiser la portée ou la dimension exceptionnelle de la famine qui provoqua entre 1932 et 1900 tu entre trois la mort de 3 5 millions d'Ukrainiens. Il pourrait être de débattre de cette qualification de génocide qui nous est proposé de voter, je l'ajoute immédiatement que je voterai ainsi que mon groupe politique, comme l'a rappelé son président Patrick Kanner. En effet, il ne nous revient pas de qualifier des faits alors que les Nations-Unies s'y sont refusés, que le débat entre historiens et pas seulement entre Russes et Ukrainiens n'est pas achevée. Non, la question n'est pas là. Et ce ne sera pas l'objet de mon propos. Une famine provoquée les par une restructuration et la confiscation de la propriété privée parfois par la constitution. De domaines coloniaux et toujours par le refus de presque tout secours aux populations abandonnées qui les conduisent à la mort l'entraîne aussi un effondrement durable de la natalité et de l'immigration. Je n'essaie dans ces conditions, mes chers collègues si l'Holodomor est ou non un génocide cette extermination par la faim et dans tous les cas un événement tragique de l'histoire universelle. Il me ramène personnellement à la plage Lytton. De lier Piazza où furent massacrés 10.000 juifs lui du ghetto de Riga. Au musée de Tuol Sleng à Phnom-Penh au musée de la mémoire et des droits humains à Santiago du Chili. Il me ramène aussi le 24 avril dernier à la commémoration du génocide de 1915 à Erevan où j'étais présent aux côtés de certains de nos collègues de tous bords politiques pour célébrer la mémoire d'un peuple en larmes et en marche qui se remémorer un génocide dont l'Europe s'est détourné. Qu'il s'agit de détruire pour soumettre ou de détruire pour éradiquer un massacre de masse répond toujours à la même logique ultime, celle de faire disparaître une population non seulement de sa terre mais de la Terre pour reprendre l'expression d'Hannah Arendt, si Massa ont par ailleurs toujours les mêmes prémisses la discrimination la persécution la marginalisation d'une communauté au regard de tous. C'est bien ce qui est commun à l'ensemble de ces événements a même processus auquel nous devons être attentifs car il est toujours à l'oeuvre. C'est pour cela que la mémoire de l'Holodomor doit être rappelé pour ce qu'il y a de l'évocation de la dimension tragique de l'histoire. Ses dimensions été excellemment évoqués par les orateurs précédents et je remercie Joëlle Garriaud-Maylam nous nous avoir permis par ce débat à la fois d'exprimer notre solidarité à l'Ukraine aujourd'hui exercer notre devoir de mémoire. C'est pour cela que le vote de cette résolution s'impose. Je vous remercie.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, mes chers collègues. Dans les années 30 une épouvantable famine a causé la mort de 7 millions de victimes civiles. Elle n'était la conséquence ni d'un dérèglement climatique ni d'un phénomène naturel d'envergure. Elle était organisée par l'homme et c'est bien, chers collègues. Un événement d'une ampleur tout à fait exceptionnel. Les victimes étaient essentiellement ukrainienne mais aussi kazakh et russe. Nous, nous demandons 90 ans plus tard. Comment qualifier ce drame avec précision et c'est la question que nous nous posons ici et aujourd'hui, je le précise pour faire écho à l'intervention de notre collègue qui est très courtoisement partie. Avons-nous le droit par respect pour les générations passées par solidarité pour ceux qui souffrent aujourd'hui par souci des générations futures de fermer encore les yeux les Européens pour la plupart ont été longtemps ignorant de cet épisode désastreux et pourtant pas si lointain dans l'histoire. Ce qui a été appelé au lieu de mort, contrairement à l'Holocauste la Shoah. N'a pas laissé beaucoup de traces dans les mémoires européenne. Il faut dire que les forces obscures de l'époque sous la forme du pouvoir en URSS ont réussi à camoufler l'horreur en 1932 une loi fut promulguée la loi des épis quelqu'un qui gardait ou caché des semences en Ukraine devenaient passibles de la peine de mort l'hiver fut glacial. Il n'y avait plus de céréales chez les paysans, plus de nourriture. La population était de plus en plus affamés elle commença par manger les animaux d'élevage et sauvages, puis les animaux domestiques. Puis les rats les racines. Certains se suicidaire enfin la population ukrainienne étant désespérée. On a même rapporté des cas d'anthropophagie. L'Ukraine de 20 alors. Un immense miroir dans l'indifférence quasi générale. Malgré des millions de morts Lénine l'avait annoncé pour soumettre un peuple, il suffit de la famille. Aujourd'hui, nous sortons d'un nouvel hiver glacial qui fait étrangement et terriblement écho à ces faits anciens confiscation approvisionnement ressources céréales populations civiles victime enfant déportation. Est-ce que les tentations génocidaires faute d'avoir été démasqués pourraient tenter de resurgir notre collègue Joëlle Garriaud-Maylam très à l'écoute du peuple ukrainien salué il y a quelques mois dans l'hémicycle par le président Rouslan Stefantchouk nous propose une excellente résolution enjoignant le gouvernement gouvernement français de reconnaître enfin le Holodomor des années 30 comme étant un génocide. Nous avons reçu madame Alexandra Matvichuk avocate ukrainienne, Prix Nobel de la paix 2022 elles-mêmes et son équipe recense des témoignages qui documente les crimes de guerre actuellement perpétrés sur le sol ukrainien de l'Holodomor. Voilà ce qu'elle dit, ce qui ne connaissent pas leur histoire sont obligés de la répéter tout le peuple ukrainien grâce à un immense courage mais aussi grâce à la certitude que le temps de la paix ne viendra pas sans le temps de la justice. Elle nous a fait comprendre avec toute son Intelligence et sa passion combien il était important pour le peuple ukrainien d'obtenir l'assurance qu'aucun Crime ne peut être dissimulée Coca ne restera impuni, que chacun d'eux sera reconnu par la communauté internationale pour ce qu'il est cher collègue les victimes de l'Holodomor nous demande la vérité. Nous leur devons et nous, nous la devons car au delà de ce drame de l'histoire en terre ukrainienne. Notre devoir est de démasquer toute volonté ou que ce soit dans le monde qu'aurait un peu plus d'infliger un autre délibérément des conditions de vie menant inexorablement à son nez anéantissement physique le le de morts était bien une intention délibérée de détruire un groupe de personnes nié son caractère génocidaire s'est grimé la mémoire des peuples. Le 26 novembre 2022, jour de commémoration Alexandra Matvichuk écrivait encore des millions de personnes sont mortes dans une terrible agonie aujourd'hui la Russie essaye d'effacer la mémoire de ce Crime la Russie démoli le mémorial aux victimes dans Marioupol occupée mais la mémoire survit et ses paroles font écho à celles du grand poète ukrainien Taras Chevtchenko notre âme ne peut pas mourir. Faisons en sorte, mes chers collègues, que notre humanité ne puisse pas mourir non plus, je vous remercie. la suite de la discussion, la parole est à monsieur Édouard Courtial pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le droit et l'espoir de l'humanité, pas la guerre. Ces mots sont ceux de Benjamin fermer le dernier procureur des tribunaux Nuremberg qui nous a quitté le 7 avril dernier. Il fut donc un acteur parmi d'eau pour que le droit prime sur la vengeance donnant ainsi malgré l'horreur et la barbarie. Une leçon aux hommes devant l'histoire et un espoir à l'humanité. Ainsi depuis 1948 les États se sont engagés conventionnellement à prévenir et punir le Crime des crimes, celui de génocide. Au sommet de l'indicible du fait de la cruauté et la barbarie qui les caractérise c'est la volonté inébranlable de faire disparaître de la surface de la Terre, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. L'adoption de cette convention est largement, le travail d'un homme un juriste polonais du nom de Raphaël Linkin. Choquée par l'impunité accordée aux responsables ottoman après le génocide arménien il dédia sa vie au combat contre le génocide, terme qu'il a d'ailleurs créé. À l'occasion d'une conférence commémorant le 20ème anniversaire de l'Holodomor Mclean a déclaré ce dont je veux vous parler. L'exemple le plus classique du génocide soviétique l'expérimentation la plus achevée en matière de russification la destruction de la nation ukrainienne. Le le de morts extermination par la faim est encore méconnu de nos compatriotes en comparaison des autres crimes de masse du 20e siècle. Cette famine organisée par le pouvoir central staliniens à partir de 32, a entraîné la mort de 4 5 à 9 millions de personnes en Ukraine. La collectivisation forcée des terrains agricoles placée sous l'autorité de Moscou. Prenons un tiers des récoltes mènent à une famine en Ukraine et malgré les alertes envoyées au pouvoir central sur la situation locale. Les directives ne feront que de se renforcer, s'apparentant à une soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, élément constitutif du génocide à l'article de. C'est de la convention de 1949. La nature génocidaire de l'Holodomor a fait déjà l'objet d'une reconnaissance entre par le Parlement ukrainien. En 2006, le parlement brésilien en 2007 encore, les parlements européen et allemand en 2022. Certaines critiques diront que la reconnaissance de ce génocide vieux maintenant de près d'un siècle au moment où la Russie envahit l'Ukraine apparaît comme une reconnaissance de circonstance. Pourtant cette reconnaissance sincère des crimes passés et rendu plus que nécessaire par les situations contemporaines. Alors que la Russie est suspecté de génocide en Ukraine avec une affaire pendante devant la Cour internationale de justice la condamnation et reconnaissance de l'Holodomor sont un signal fort de solidarité et de la position de la France qui combattra toujours l'impunité des criminels internationaux. comme la reconnaissance du génocide arménien toujours nié par la Turquie la réalité historique de l'Holodomor est aujourd'hui encore plus qu'hier, ni par la Russie. L'adoption de cette résolution est donc un moyen pour la France de s'élever et de relayer la voix des victimes et de l'Ukraine. Face au choix de la Russie du Ilon c'est du révisionnisme cette résolution encourage à ouvrir un travail de fond de réflexion historique et mémoriel juste et indispensable et je tiens donc à saluer cette initiative portée par notre collègue Joël Guerriau mais. Que je vais bien évidemment soutenir. Car si on ne veut répéter les erreurs du passé et ne pas être aveugle à celle du présent ah regard juste de l'histoire est nécessaire. Qualifié l'Holodomor de génocide, c'est reconnaître une réalité immuable. Merci. Merci cher collègue. Pour terminer cette discussion générale. La parole est à monsieur Olivier Becht, Ministre délégué chargé du commerce extérieur de l'attractivité et des Français de l'étranger. Merci beaucoup monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs. Céline. La résolution que le sénat examine aujourd'hui revêt une importance toute particulière. Non seulement parce que la mémoire de la grande famine ukrainienne de 1932, 1933 10 le de morts est devenue un élément central de l'identité du pays. Mais aussi parce que les souffrances alors endurées par le peuple ukrainien font écho à celles qu'il subit aujourd'hui. Alors que la capitale Kiev a encore été visées hier par des missiles hypersoniques russes. D'hier à aujourd'hui, en effet, la détermination dans la nation ukrainienne fait preuve au cours de l'histoire forcent notre admiration. Ce texte est également important car il souligne l'envergure de ce Crime de masse qui est le lot de morts resté longtemps méconnu en raison de la volonté des autorités soviétiques de dissimuler les preuves attestant de leur implication dans son organisation. Il a ainsi fallu attendre l'arrivée au pouvoir de Monsieur Gorbatchev, pour que la vérité se fasse progressivement jour grâce au travail des historiens qui à partir de l'exploitation des archives ont mis en le mis en lumière les réalités du projet soviétique. Celui-ci ne visait rien moins que l'écrasement d'un ennemi intérieur fantasmer. Le Coulac. Paysan possédant que le régime considéré également comme le représentant d'un nationalisme ukrainien cherchant à saboter sa politique de collectivisation forcée. Pour atteindre ce but, le régime a recouru aux amandes oh confiscation des moindres réserves de nourriture mais aussi au blocus du village entier fuyant la famine et enfin aux déportations collectives. Cette répression implacable, a fait plusieurs millions de morts. La résolution que vous examinez aujourd'hui revêt une signification toute particulière. En raison de sa résonance évidente avec l'actualité. La Russie cherche aujourd'hui à instrumentaliser l'histoire. Afin de nourrir un récit national, justifiant ses ambitions impérialistes et sa guerre d'agression contre l'Ukraine. Elle pousse la manipulation des événements jusqu'à la dénégation de la réalité de l'Ukraine comme peuple et comme nation. Face à ces agissements. La France poursuit son soutien au travail indispensable des historiens. commissions pardon programme que nos unités mixtes de recherche en France et à l'étranger ont mis en place avec l'Ukraine en histoire et en sciences sociales, l'attachement à la vérité des faits historiques. Et la marque et des nations démocratiques. La dernière commémorations de l'Holodomor le 26 novembre dernier a rappelé avec une acuité toute particulière que la Russie aggrave par. Et la guerre d'invasion. L'insécurité alimentaire mondiale dont de nombreux États souffre aujourd'hui. Là encore, la France a agit avec résolution. Le président de la République, il avait annoncé à cette occasion le soutien de la France à l'initiative Green from Ukraine lancée par le président Zelensky qui c'était très concrètement traduit par une contribution supplémentaire de 6 millions d'euros pour le transport et la distribution par le Programme alimentaire mondial de céréales d'Ukraine à destination du Yémen et du Soudan. À travers cette proposition de résolution. Vous vous inscrivez dans ce travail de reconnaissance d'un crime indéniable. Comme l'a fait. L'Assemblée nationale il y a peu et d'autres parlements à travers le monde. Comme je l'avais indiqué lors de l'examen à l'Assemblée nationale, il n'est pas dans les habitudes du gouvernement de reconnaître comme génocide des faits qui n'ont pas préalablement été qualifiés comme tels par une juridiction qu'elle soit française ou internationale. Mais la réalité des crimes commis lors de l'eau de morts ne fait pas de doute. Et c'est pourquoi le gouvernement soutient ce texte. Je tiens à redire ici le soutien. Constant indéfectible, monsieur l'ambassadeur. De la France à l'Ukraine. Pour l'aide à se défendre mais également l'aide à tenir. C'est ce message qu'il a passé le président de la République au président Zelensky ce dimanche encore pour le 2ème déplacement de ce dernier dans notre pays depuis le déclenchement de l'agression. Au delà des nouvelles livraisons d'équipements militaires notre soutien vient répondre à l'ensemble des besoins exprimés. Aide économique et financière. Aide humanitaire et aide matérielle, lutte contre l'impunité. Au total, le soutien de l'Union européenne des ses membres dépasse les 67 milliards d'euros. En défendant l'Ukraine dans cette guerre d'agression. La France et l'Union européenne défendent également l'idée d'un ordre international basé sur le droit et sur les règles. Face à la Russie de plus en plus isolé y a dont le président est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et qui ne montre aucune ouverture pour la négociation et le dialogue, le soutien à l'Ukraine et la seule option. Car, aider l'Ukraine à résister et à reprendre l'ascendant et la meilleure manière de mettre un terme au conflit. La France agit donc concrètement pour ne pas laisser les crimes du passé sous silence. Pas plus qu'elle ne tolère l'impunité de ceux aujourd'hui commis par la Russie sur le sol ukrainien. C'est le message qu'ont rappelé le président de la République et la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères lors de leurs interventions respectives au sommet de Boutcha, 31 mars et au sommet du kangourou sur l'établissement d'un tribunal spécial pour juger les crimes d'agression. C'était le 9 mai dernier. C'est tout le sens de notre appui concret continue aux autorités ukrainiennes en matière de lutte contre l'impunité. Nous leur avons remis le 9 mai un 2ème laboratoire d'analyse ADN qui permettra d'appuyer les enquêtes menées par les juridictions ukrainienne et de participer à la documentation des crimes commis dans le cadre de l'agression russe. Nous continuerons à agir en ce sens aux côtés de l'Ukraine. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Ministre, nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution, la conférence des présidents, a décidé que les interventions des orateurs Valais. Explications de vote. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur l'ensemble de la proposition de résolution. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées que 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 343 exprimés, 343 pour 327 contre 16, le Sénat a adopté. Mes chers Mes chers collègues. Je vais suspendre la séance. Prochaine séance. Je pense mardi. Mardi 23 mai à 14h 30 pour les explications de vote, des groupes puis de scrutin public sur sur la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France. La séance est levée.